pour le groupe La République En Marche.

le débat sur la mise en oeuvre ambitieuse par le Gouvernement du reste à charge zéro a été relancé il y a quelques jours après qu'une

la décision de la Cour de cassation donnant raison à la crèche Baby-Loup contre une salariée licenciée en 2008 pour non-respect du règlement intérieur. Le 23 octobre dernier, il a rendu un nouvel avis

à la fois la dignité de toute personne et le respect de l'ordre public dans sa dimension de sécurité. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, avait jugé que cette loi ne portait atteinte ni à la liberté de conscience ni à la liberté religieuse, et qu'elle n'était en aucun cas discriminatoire.

ce comité demande des comptes à la France, sans pour autant en demander aux pays qui violent des droits humains les plus élémentaires dans le plus grand silence. Ses invectives à répétition sont inquiétantes, laissant croire au monde entier qu'il a un pouvoir juridictionnel. Or seules les juridictions européennes et françaises sont compétentes, et elles se sont déjà prononcées sur notre législation avec l'autorité de la chose jugée. Le Gouvernement ne doit pas faiblir face à ce qui relève d'un véritable parti pris idéologique. Madame la garde des sceaux, demain 26 octobre se tiendra l'assemblée générale des Nations unies. Le 10 décembre, nous célébrerons le soixante-dixième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme

ce comité a estimé que l'interdiction de porter le voile intégral en public constituait une atteinte disproportionnée au droit des deux plaignantes de librement manifester leur religion.

que la loi de 2010 apportait une conciliation équilibrée entre liberté religieuse et protection de l'ordre public. La Cour européenne des droits de l'homme elle-même en formation plénière a estimé en 2014 que cette loi était conforme dans la mesure où la préservation des conditions du vivre ensemble était un objectif légitime, qui permettait d'interdire le voile intégral.

et plus respectueuse de chacun. Bien sûr, toute personne est libre de porter dans l'espace public un vêtement destiné à manifester une conviction religieuse. Toutefois, la loi peut interdire la dissimulation du visage, dans la mesure où cela est jugé incompatible avec les principes de sécurité et de fraternité qui fondent la société démocratique dans laquelle nous vivons. La parole est

Il y a dix mois, à l'occasion du, votre collègue ministre de l'économie et des finances promettait que « désormais, chaque euro placé dans un livret de développement durable et solidaire- LDDS -centralisé à la Caisse des dépôts sera[it] associé à un projet contribuant effectivement à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique de notre modèle économique ». C'est un engagement très fort.

En effet, le fonds d'épargne qui gère 60 % des 100 milliards d'euros d'encours épargnés au titre du LDDS est actionnaire d'entreprises pétrolières, minières ou automobiles : un comble ! montant, seulement 10 milliards d'euros sont effectivement consacrés à la transition énergétique, et encore uniquement à la rénovation thermique du bâti ancien, seul cas de figure prévu par la loi. Pis encore, nous n'avons aucune information, ou presque, sur les 40 milliards d'euros gérés directement par les banques. Elles doivent pourtant publier un rapport annuel précisant l'utilisation de cette épargne. Cette publication indigente, que l'on n'ose appeler « rapport », tient en une page. Pourquoi diable exclure Pourquoi diable exclure ces fonds du champ d'action ? Chaque épargnant doit être informé de manière détaillée de l'utilisation de son argent. Soyons clairs avec les 24 millions de Français détenteurs d'un très mal nommé livret de développement durable non seulement leur argent finance très peu la transition écologique, mais il finance parfois le réchauffement climatique ! Le défi à relever par le Gouvernement est donc colossal. Il faudrait changer la loi pour inclure dans le dispositif le financement de toute la transition énergétique, notamment les collectivités locales. Il faudrait également contrôler drastiquement les activités boursières du fonds d'épargne et répondre favorablement à l'interpellation d'ATTAC. Et conclure ! Monsieur le ministre d'État,

la collecte du livret de développement durable et solidaire centralisée au sein du fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations sera affectée au financement de projets ayant un impact positif sur le climat.

La centralisation de ces dépôts a ainsi permis au fonds d'épargne de financer ce secteur à hauteur de 160 milliards d'euros, tandis que les actifs financiers qu'il détient- ce ne sont pas que des actions, il y a également des obligations, par exemple -, qui ont vocation à assurer sa liquidité, sont gérés selon les principes de l'investissement responsable au regard de la transition écologique et énergétique.

La disparition, le 2 octobre dernier, du journaliste d'origine turque Jamal Khashoggi a déclenché une véritable onde de choc dans le monde. Il y a tout d'abord les conditions de cette disparition : au sein du consulat saoudien à Istanbul et, si l'on en croit le président turc Erdogan, il s'agirait d'un assassinat particulièrement sordide. Au-delà de ces circonstances et de cette brutalité qui choquent, il ne s'agit pas simplement d'un fait divers. J'en veux pour preuve l'adresse du président Erdogan au parlement turc, les déclarations du président Trump, celles des responsables européens, le retrait d'un certain nombre de grands investisseurs du monde entier du sommet de Riyad, mais aussi le déplacement plus discret de la directrice de la CIA en Turquie et les rencontres entre Mohammad ben Salmane, personnage central de cette affaire,

La chancelière allemande appelle à cesser l'exportation des armes vers l'Arabie saoudite, qui -faut-il le rappeler ? -conduit une guerre meurtrière au Yémen. Comment la France, qui depuis 2008 a exporté pour 11 milliards d'euros d'armes en Arabie saoudite, considère-t-elle cette déclaration de l'Allemagne ? Quelques mois avant les élections au Parlement européen, l'Europe ne donne-t-elle pas une image de plus de sa désunion ? Plus largement, car on voit bien que cette affaire dépasse ses protagonistes, comment notre pays voit-il la sortie de ce qui pourrait être une crise déstabilisatrice ? La Turquie, héritière de l'Empire ottoman, n'est-elle pas en train de faire monter la pression en distillant les informations à petites doses ? Que cherche-t-elle à obtenir des Américains, des Saoudiens ? La domination du monde musulman sunnite, par le rétablissement du califat ? La ne va-t-elle pas finalement reprendre le dessus, les importations de pétrole saoudien et les exportations d'armement valant bien plus que la vie d'un homme que l'on dit par ailleurs proche des Frères musulmans et de Ben Laden ?

Vous l'avez fort bien rappelé, il s'agit, avec l'affaire Khashoggi, du meurtre, dans une enceinte diplomatique, d'un journaliste saoudien contributeur régulier à la presse internationale.

juste titre l'indignation de la communauté internationale et appelle, de la part des autorités saoudiennes, une réponse transparente et exhaustive. C'est ce que la France et ses partenaires ont demandé à l'Arabie saoudite. C'est l'objet de nos entretiens avec nos homologues saoudiens à tous les niveaux, y compris entre le Président de la République et le roi Salmane, hier, et entre le ministre des affaires étrangères et les autorités saoudiennes. Les autorités saoudiennes ont reconnu le caractère de « meurtre » s'attachant à la mort de M. Khashoggi. Cependant, elles n'ont pas encore, à ce jour, établi les circonstances exactes de cette mort ni les responsabilités engagées. La France demande que les enquêtes qui sont diligentées fassent toute la lumière sur la manière dont un tel meurtre a pu être commis. Nous l'attendons de l'Arabie saoudite. Nous avons avec ce pays une relation politique et stratégique forte, fondée sur des intérêts communs, qui crée aussi des attentes, notamment en matière de respect des droits de l'homme : nous vérifierons qu'elles sont bien prises en compte. Nous le devons d'abord à la famille et aux proches de M. Khashoggi.

Je suis convaincu que, dans les deux cas, tous les services publics concernés, spécialement la marine nationale en Méditerranée, ont fait leurs meilleurs efforts. Pour avertir et donc prévenir, tout d'abord : dans un cas, l'alerte aux navires a été lancée par le CROSS, le

des agents publics et des bénévoles pour lutter contre la pollution. Nous prenons des mesures supplémentaires et, s'il le faut, nous agirons pour modifier le droit maritime international afin de mieux protéger les populations contre ces risques.

Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. La suppression de la taxe d'habitation, que personne n'a demandée, représenterait un manque à gagner de 26,3 milliards d'euros en 2020. Le Gouvernement reprend dans le même temps cet argent aux Français en créant et en augmentant d'autres taxes, qui affectent la grande majorité de nos concitoyens : annonce de la création de la vignette poids lourds, hausse de la fiscalité dite écologique par le relèvement de la taxe sur les carburants-

monsieur le Premier ministre, c'est beaucoup trop pour la très grande majorité de nos concitoyens, qui ont besoin d'utiliser leur véhicule au quotidien, tout simplement pour vivre et travailler. En un an, le prix du gazole a augmenté de 25 %.

La France est l'un des pays occidentaux les moins pollueurs, mais les Français sont parmi les plus taxés. L'impôt est efficace quand il est juste. Les Français sont saturés de la fiscalité « verte » car elle devient punitive Monsieur le Premier ministre, les Français n'en peuvent plus : quand allez-vous réellement faire des économies au niveau du fonctionnement de l'État et en finir avec ces hausses et créations de taxes ?

une grande partie du territoire souffre d'une sécheresse persistante. Ce phénomène climatique de grande ampleur a des conséquences multiples, telles que d'importants mouvements de terrain provoquant des fissures impressionnantes sur nombre de constructions. La sécheresse est également dramatique pour nos agriculteurs et nos éleveurs. Les éleveurs, notamment, n'ont plus de trésorerie, et la saison prochaine est déjà compromise.

de retenir le principe d'un dégrèvement collectif de la taxe sur le foncier non bâti à hauteur des taux de pertes fourragères, établis par les comités d'expertise des calamités agricoles. Monsieur le ministre, ma question est simple : le Gouvernement est-il prêt à entendre ces demandes, qui ne visent, au demeurant, qu'à la juste réparation d'un préjudice certain ?

Les volontés précaires se traduisent par des discours, les volontés fortes par des actes. » À bientôt, monsieur le ministre ! La parole est à M. Bernard Cazeau, pour le groupe La République En Marche. Ma question

Pour autant, sur le terrain, nombre de réorganisations industrielles en cours méritent une attention spécifique des pouvoirs publics, notamment celles qui relèvent essentiellement du coût de l'énergie. Il en va ainsi des papeteries de Condat, en Dordogne. Premier employeur privé du département, ce site industriel moderne produit annuellement plus de 400 000 tonnes de papier couché de grande qualité et emploie plus de 500 salariés. Il réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 300 millions d'euros.

décision fut prise sans se référer aux politiques publiques d'aides menées par nos voisins en Europe. Récemment, un projet de chaudière biomasse présenté par l'entreprise n'a pas été retenu par l'État au titre des aides directes à la production énergétique. Aujourd'hui, il est nécessaire que la transition énergétique de cette entreprise soit accompagnée, d'autant qu'elle veut mettre en oeuvre, sur l'une de ses lignes de production, un projet industriel parallèle plus rentable, qui lui permettra de résoudre l'équation de sa compétitivité à moyen et long termes. Monsieur le ministre d'État, c'est aujourd'hui l'ensemble du bassin économique du Terrassonnais et, plus globalement, du Périgord qui attend de votre part une action à la mesure de la gravité de l'enjeu.

L'appel d'offres de cogénération par la biomasse que l'État a lancé en 2016 n'a pu aboutir, car les solutions qui ont été présentées se sont révélées beaucoup trop chères pour le budget de l'État. Nous privilégions désormais plutôt la biomasse pour la génération de chaleur.

La justice a accordé à Ascoval, placée en redressement judiciaire, deux semaines de sursis supplémentaires pour trouver un repreneur. Il ne faudrait pas que ce soient deux semaines pour rien Le groupe Vallourec, qui détient 40 % de l'usine, refuse d'apporter le soutien financier demandé par Altifort, candidat à la reprise. Or, sans Vallourec, personne n'accepte de s'engager.

Toute politique industrielle en France est-elle abandonnée au profit de la, un modèle qui promeut le chacun pour soi ?

vous m'interrogez sur la politique industrielle du Gouvernement et le devenir du site Ascoval. Permettez-moi d'abord d'adopter une perspective large, pour rappeler quelques éléments factuels.

que l'investissement poursuit sa progression- de l'ordre de 3,1 % par an en moyenne sur les cinq dernières années. Et alors ? Notre politique industrielle est avant tout une politique de reconquête industrielle pour créer les emplois de demain. Il ne s'agit pas que de la que vous avez évoquée cela passe par l'accompagnement de la transformation numérique des entreprises industrielles. Financer l'impression 3D ou encore les robots à commande numérique, c'est préparer Ce projet est étayé par un plan de 500 millions d'euros dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, avec l'octroi d'un suramortissement pour l'investissement dans les machines de l'industrie du futur.

Vallourec 2 800 emplois en France. Vallourec a perdu 300 millions d'euros au premier semestre. Il convient d'aborder ce dossier de manière responsable, de s'assurer que le seul projet de reprise qui soit aujourd'hui sur la table après que l'État a approché plus d'une centaine de repreneurs route. Je constate que, dans ce dossier, le repreneur entend investir 10 millions d'euros, alors qu'il y a plus de 150 millions d'euros à financer. Je rappelle

ont débouché sur une libération de la parole des professeurs, au travers de la campagne #PasDeVague. « Pas de vague », depuis des années, c'est l'injonction adressée à des professeurs bâillonnés par une hiérarchie paralysée par la peur du scandale. Pas de vague », c'est la seule réponse donnée aux enseignants confrontés aux incivilités, aux insultes et aux violences. Il aura fallu la diffusion sur internet d'une vidéo pour que les professeurs commencent à être entendus. Vous qui vous présentez comme le « ministre des professeurs », vous qui parlez d'« école du respect », vous ne pouvez plus tolérer, comme ce fut longtemps prôné, que la parole de l'élève vaille celle du maître, que ce soit uniquement au maître de respecter l'élève, que le concept d'autorité soit relativisé au sein même de l'école. Désormais, il faut des actes. Quels moyens humains et quel arsenal de sanctions comptez-vous donner aux chefs d'établissement ? Comment comptez-vous agir pour redonner confiance à des professeurs démoralisés et rendre le métier de nouveau attractif ? Allez-vous enfin enterrer une école de pensée qui, de Bourdieu à Meirieu, a fini par affaiblir gravement l'école de la République ? Monsieur le ministre, depuis que vous êtes arrivé au Gouvernement, la parole a évolué. Mais il est désormais temps que, sur le terrain, les professeurs, les parents, les élèves voient un changement et qu'un terme soit mis à un laxisme qui n'a que trop duré

Comme si cela ne suffisait pas, monsieur le ministre, vous défendez, au travers du projet de loi de finances pour 2019, la suppression du taux réduit pour la taxe sur le gazole non routier.

Disons-le très franchement, les grosses entreprises survivront toujours. Mais des plus petites ? Ce sont elles qui emploient le plus de salariés dans la plupart des territoires, tel mon département, l'Aveyron. Eh oui, monsieur le ministre, l'artisanat est la première entreprise de France ! Ses entreprises font vivre des populations qui habitent nos départements et qui consomment sur place. C'est tout un tissu économique local, qui représente beaucoup d'emplois non délocalisables.

Sans solutions anticipées, le rétablissement des barrières douanières et des formalités requises pour le transit des produits phytosanitaires ou d'origine animale risque d'entraver fortement la circulation des marchandises. La rapidité et la simplicité des démarches administratives sont essentielles pour fluidifier le trafic et garantir un modèle économique portuaire concurrentiel. Après l'entrée en vigueur du Brexit, le Royaume-Uni sera considéré comme un pays tiers. Toutes les marchandises en sa provenance seront soumises à des contrôles douaniers. Les produits phytosanitaires et d'origine animale feront, en outre, l'objet d'une procédure de déclaration spécifique. Ces formalités mobiliseront des personnels des services vétérinaires et phytosanitaires supplémentaires. L'alourdissement des formalités, l'allongement des délais et la mobilisation d'espace foncier vont peser fortement sur l'équilibre économique du transport des marchandises. Sans anticipation, les ports normands, comme ceux du Havre et de Dieppe, seront fortement touchés. Ma question est simple : quelles mesures le Gouvernement entend-il adopter pour faciliter les échanges maritimes, notamment pour les produits phytosanitaires et d'origine animale ? Comment compte-t-il financer les investissements nécessaires à la mise en oeuvre de ces nouvelles procédures ?

sénatrice Canayer, les discussions entre le négociateur européen et le Royaume-Uni n'ont malheureusement pas permis, à ce stade, d'aboutir à un accord sur l'ensemble des modalités de retrait du Royaume-Uni

et, en même temps, de ne pas porter atteinte à l'intégrité du marché unique européen. Cette solution doit encore être trouvée avec les Britanniques, qui, pour l'heure, ont rejeté les propositions européennes. Dans ce contexte, les chefs d'État et de Gouvernement ont réaffirmé leur confiance dans le négociateur européen, leur volonté de rester unis dans cette négociation et la pertinence du mandat donné à Michel Barnier. Cette solidité de l'ensemble des partenaires européens sur un sujet aussi important est précieuse. Ils ont indiqué, en outre, qu'un conseil européen extraordinaire pourrait être convoqué à tout moment si des progrès décisifs étaient réalisés avant le conseil européen du mois

la solution doit être trouvée très rapidement. Des choix politiques lourds doivent être opérés par les autorités britanniques. Les incertitudes qui pèsent sur l'issue des négociations soulignent plus que jamais la nécessité de nous préparer à toutes les éventualités, y compris celle de l'absence d'un accord

Compte tenu des contraintes budgétaires qui pèsent sur l'État et les collectivités territoriales, le recours à une combinaison de financements publics et privés est devenu indispensable pour assurer la pérennité des projets culturels et éviter que leurs acteurs ne soient trop exposés aux conséquences brutales du retrait de certains de leurs financeurs. C'est vrai pour le spectacle vivant, les arts plastiques, les musées, ainsi que pour la préservation du patrimoine, domaine dans lequel les besoins de financement sont particulièrement criants, comme en témoignent les conclusions de la mission confiée par le Président de la République à Stéphane Bern il y a quelques mois.

aurait pu constituer un premier coup de canif à la loi Aillagon, laquelle n'a jamais été remise en cause depuis son adoption en 2003. Le signal aurait été d'autant plus négatif que, après les dernières réformes fiscales- je pense en particulier au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et, immobilière -, les associations et fondations ont déjà enregistré une baisse drastique du montant des dons qui leur sont consentis. Certes, il ne faut jamais oublier que, au-delà de la générosité des mécènes, l'État est bien le principal contributeur des actions de mécénat, par la perte de recettes fiscales à laquelle il consent. Mais, compte tenu des bienfaits manifestes de ce mécanisme pour l'intérêt général, est-il vraiment opportun de vouloir y porter atteinte ? Jean-Jacques Aillagon, que j'ai auditionné dans le cadre de notre mission d'information, en mai dernier, a lui-même déclaré, paraphrasant Montesquieu, qu'il ne fallait y toucher que d'une main tremblante. Je sais que le ministre de l'action et des comptes publics s'est engagé à ce que le Gouvernement dépose un amendement à la seconde partie du projet de loi de finances tendant à relever le plafond pour les TPE, comme nous l'avions préconisé, et à autoriser une évaluation du dispositif, ... Il faut conclure ! ...afin de détecter les cas éventuels d'« optimisation aggravée le ministre, quelle est la position du ministère de la culture sur ce dispositif fiscal, créé et défendu par l'un de vos prédécesseurs ? Comment entendez-vous garantir le respect des engagements pris par le Président de la République, tant à l'Élysée que lors de son déplacement dans les Yvelines ?

C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a demandé à la Cour des comptes un rapport, qui sera remis prochainement. Les conclusions de ce rapport devront être étudiées par les

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, toutes les initiatives parlementaires relatives aux droits des aidants convergent depuis plusieurs mois. Elles visent à reconnaître l'engagement d'une population qui assume à elle seule une action médico-sociale invisible, venant en déduction de la charge de l'État. Ces démarches sont à chaque fois transpartisanes

cette initiative, nous souhaitons relever le défi de la prise en compte des aidants par la Nation, dans sa dimension tant publique que privée. Lors de mes travaux préparatoires, une question s'est imposée

Les dispositifs d'aide et d'information manquent de rationalité. L'État ne tient malheureusement pas sa place. Son action manque de coordination et de proactivité envers ceux qui lui font pourtant économiser jusqu'à 16 milliards d'euros par an. Les aidants sont susceptibles d'entrer dans un isolement profond, voire une détresse dangereuse. Nous partageons tous cette responsabilité. J'ai reçu de nombreux témoignages, notamment celui d'une mère dont l'enfant est atteinte d'une maladie rare. Cette enfant qui ne dort presque jamais, ne s'exprime qu'en criant et s'agite en permanence ne peut pas être prise en charge, tant sa pathologie est lourde, exigeant une assistance de chaque instant. N'en pouvant plus, isolée bien qu'épaulée par son conjoint, sa mère a failli. Elle a attenté à la vie de sa fille en lui administrant trop de médicaments. Aujourd'hui, la personne la plus experte pour s'occuper de cette enfant est séparée d'elle. La famille est détruite en raison du manque de soutien et de l'isolement créé par cette situation. situation. Je ne peux m'empêcher de penser à ma soeur et à mon beau-frère, qui ont élevé leur fille Léa, atteinte du syndrome de Rett : quel n'a pas été leur épuisement physique, mais aussi psychologique Ces vies sont celles de nombreux Français. Malheureusement, nous avons tous, autour de nous, un exemple de ce type. Nous ne pouvons pas ignorer ces situations. La question est donc simple : qui doit s'occuper des aidants ? La réponse est : nous, Parlement et Gouvernement, maintenant ! La réponse est : la société. La réponse est : chacun d'entre nous.

Il eût été aisé de s'en remettre à lui pour trouver les moyens de financer ces actions. Mais les mesures innovantes que nous proposons ont une valeur thérapeutique pour celles et ceux que l'on oublie, qui souffrent, qui s'isolent, et qui parfois même décèdent avant la personne qu'ils aident.

Je ne doute pas que le Gouvernement serait arrivé, et arrivera, aux mêmes conclusions. Je salue l'excellent travail de notre rapporteur, M. Olivier Henno. Il a parachevé l'ouvrage que j'ai tissé au cours des derniers mois,

C'est donc après un travail collaboratif et approfondi que la commission a modifié utilement certaines mesures, tout en partageant les objectifs que je m'étais fixés. Ainsi, l'indemnisation du congé de proche aidant, financée par un fonds privé, ne crée pas de charges supplémentaires ou nouvelles pour l'État.

Pour répondre à cet enjeu, nous proposons d'assurer l'identification de l'aidant et de renforcer sa reconnaissance par le corps médical. Il s'agit de le détecter pour l'informer rapidement de ses droits, pour le mettre en contact avec les bons interlocuteurs et en lien avec les réseaux associatifs.

Les salariés deviennent parfois des aidants, et l'on ne saurait considérer qu'il s'agit là d'un choix de leur part. C'est pourquoi les branches professionnelles devront étudier les possibilités de coordination et de souplesse entre la vie personnelle de l'aidant et sa vie professionnelle. Cette disposition, soutenue par Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail, a été adoptée lors de l'examen du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, mais le Conseil constitutionnel l'a censurée, considérant qu'elle constituait un cavalier législatif. Ici, elle a toute sa place. permettre l'indemnisation du congé de proche aidant, notre solution est novatrice. L'État ne déboursera pas un centime- une fois n'est pas coutume -, et l'exécutif devrait s'en saisir Notons bien qu'il s'agit non pas d'une professionnalisation de l'aidant, mais d'une compensation de la perte de salaire qu'il subit en prenant ce congé. Ce dispositif est parfaitement expliqué dans le rapport. Accepter le principe de la mise en place d'une surcote pour certains contrats d'assurance est sans aucun doute un choix politique. Pour ma part, je considère que, le taux étant faible, il peut totalement être assumé, à l'instar de l'éco-participation, par exemple. Madame la secrétaire d'État, je ne souhaite pas que nous adoptions un simple texte d'affichage. J'ai le désir que nos travaux aboutissent à une rédaction compatible avec l'agenda du Gouvernement, en particulier pour l'harmonisation des droits sociaux des aidants.

À la demande du Président de la République, les travaux consacrés à la dépendance se sont ouverts avec le chantier « grand âge et autonomie » lancé le 1 octobre dernier. Un atelier aborde la question des aidants. Nos propositions ne vident certainement pas le sujet, notamment du fait de l'application de l'article 40 et des échanges qui doivent avoir lieu entre ministères.

ou encore à la faculté, pour les aidants, de cumuler des droits à la formation : on sait que le retour à l'emploi est extrêmement compliqué pour ce public. Nous serons attentifs

Or ce sujet connu de longue date exige une réponse ; il faut agir dès maintenant. Les solutions connues aux demandes identifiées ne changeront pas d'ici à 2019.

J'invite donc le Gouvernement à se saisir de ce véhicule législatif, à poursuivre ses travaux pour en consolider et enrichir le dispositif par la suite. Attendre, c'est faire peser un poids chaque jour plus insupportable sur les épaules des aidants. Madame la secrétaire d'État, voilà plusieurs mois que l'on joue, au Parlement, une douce et tenace mélodie au sujet des aidants, de leurs droits et des aides qui peuvent leur être apportées. Aujourd'hui, nous avons un devoir de résultat. Nous avons même un devoir humain : celui d'engager une action, de sécuriser ceux qui donnent gratuitement de leur temps, qui donnent gratuitement une part de leur vie. Le dispositif de cette proposition de loi repose sur le bon sens et l'innovation. J'ajouterai qu'il y a surtout des réponses, mais que, plus encore, il y a l'État ; l'État qui accompagne, l'État qui n'ignore pas, l'État qui soutient.

N'oublions pas que l'on juge un État à sa manière de traiter les anciens et,, les personnes handicapées ou dépendantes. Aujourd'hui, les aidants supportent une partie de la charge qui incombe à l'État. Nous avons une dette C'est donc avec la plus profonde conviction que j'apporterai mon soutien au texte tel que présenté par M. le rapporteur. Mes chers collègues, je vous invite à suivre cette voie, et j'espère que l'Assemblée nationale pourra prochainement se prononcer sur ce texte, pour apporter enfin des réponses à une population sans laquelle la France ne serait pas à la hauteur de ses prétentions ! La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, nous voici réunis pour l'examen d'un texte dont la Haute Assemblée a toutes les raisons de s'enorgueillir.

physiques. Cette mauvaise santé des aidants interpelle encore trop peu le personnel soignant ou les équipes médicales. Ainsi, seuls 13 % des aidants affirment être interrogés sur leur santé quand ils accompagnent leur proche aidé à l'hôpital.

Voilà un texte qui s'inscrit dans le droit fil d'un engagement parlementaire en faveur des aidants qui ne se dément pas depuis plus de deux ans. Directement inspiré du rapport de notre collègue Jocelyne Guidez sur la proposition de loi ouvrant la possibilité de faire don de jours de repos non pris à un collègue proche aidant, ce texte se réclame également de la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par notre collègue député Pierre Dharréville et de celle qui a été très récemment déposée au Sénat par nos collègues du groupe CRCE. De tous les horizons politiques de nos deux assemblées, c'est un mouvement spontané et uniforme qui émerge progressivement pour se saisir d'une question urgente, n'ayant été jusqu'à présent qu'imparfaitement et indirectement traitée.

À l'évidence, nos intentions sont partagées, mais nous sommes poliment invités par le Gouvernement à les contenir. Faut-il attendre que la réforme de la prise en charge de la dépendance, la réforme des retraites et l'évolution de l'accompagnement des personnes handicapées intègrent un volet relatif aux aidants ?

et, surtout, disparate. Entre les retraites, la dépendance, l'évolution quinquennale de l'accompagnement du handicap et la stratégie nationale pour l'autisme, ce sont pas moins de quatre grands chantiers dont la feuille de route prévoit un volet relatif aux aidants.

un sujet à part entière. Les chiffres sont désormais connus : plus de 8 millions de personnes se consacrent quotidiennement à l'accompagnement d'un proche, dont la perte d'autonomie, qu'elle soit liée à l'âge ou à un handicap, rend nécessaires une présence et une surveillance continues. Bien qu'aucune d'entre elles ne réclame la création d'un statut, d'un droit à part, elles sortent peu à peu de la discrétion à laquelle leur mission et le faible soutien des pouvoirs publics les contraignent souvent. Mes chers collègues, nous savons qu'il n'est plus possible de considérer l'accompagnement du proche aidé comme une simple extension de la solidarité familiale ; c'est une mission qui se situe entre le métier et le devoir, sans se confondre avec aucun des deux. C'est pourquoi il est troublant que cette mission n'ait jamais été prise en compte par les politiques de solidarité nationale, dont elle relève pourtant. Ce texte apporte un début de réponse. Il embrasse très largement l'ensemble des droits sociaux des aidants et vise à assurer à ces derniers une sécurité financière

C'est pourquoi nous avons voulu instaurer l'indemnisation du congé de proche aidant : c'est le coeur de notre proposition de loi. De plus, ce texte corrige plusieurs iniquités de droits entre proches aidants d'une personne âgée et proches aidants d'une personne handicapée. Enfin, il prévoit une amélioration substantielle des modalités d'information de l'aidant et le renforcement de sa place dans le parcours de la personne qu'il accompagne. Pour conclure, je me félicite de ce que notre commission des affaires sociales ait salué l'initiative de notre collègue et adopté un texte équilibré et abouti. Mes chers collègues, ce sujet fait consensus dans l'opinion ; il n'est plus temps d'attendre. La cause des aidants est grande parce qu'elle a sa part d'humanité et de solidarité. Les proches aidants nous parlent et nous rappellent, à la suite de Jacques Delors, que, en matière de solidarité, ce sont souvent les plus fragiles qui sont les plus grands. La parole

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, madame Jocelyne Guidez, permettez-moi tout d'abord de rappeler l'importance que le Gouvernement accorde à la question des proches aidants. Le soutien aux proches aidants était un engagement de campagne du Président de la République. À ce À ce titre, il figure dans la feuille de route confiée par le Premier ministre à Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, ainsi qu'à Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Il s'agit de prendre en main une question de société qui nous concerne tous : nous connaissons tous des aidants d'un parent âgé, d'un enfant en situation de handicap, d'un conjoint malade. Certains d'entre nous sont eux-mêmes aidants, ou auront peut-être besoin un jour d'un aidant. Il faut donc saluer le dévouement exemplaire de ces millions d'aidants, signe que la solidarité est une valeur très forte dans notre société. Le vieillissement de la population renforcera le rôle fondamental des proches aidants à l'avenir. Cela doit nous conduire à nous interroger sur le soutien que nous voulons et que nous devons apporter à nos aidants. Comment les soutenir au quotidien dans leur action d'aidant ? Comment préserver leur santé, leur vie professionnelle quand ils sont encore actifs, ainsi que leur vie sociale ? Je sais que ce sont les préoccupations qui vous guident, et je salue la volonté de la Haute Assemblée de prendre ce sujet à bras-le-corps, volonté qui se traduit aujourd'hui par l'examen de la proposition de loi de Mme la sénatrice Jocelyne Guidez. Depuis près d'un an maintenant, les initiatives parlementaires de tout bord en faveur des proches aidants se multiplient, avec des propositions de loi ou des amendements à de nombreux projets de loi. Le Gouvernement se félicite de cette volonté commune, transpartisane d'avancer sur ce sujet de société. Beaucoup de choses ont déjà été faites en faveur des proches aidants. La loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement apporte indéniablement des avancées majeures, notamment par la création du congé de proche aidant ou encore la consécration d'un droit au répit des aidants. Plus récemment, le Gouvernement a souhaité diversifier les solutions de répit en s'inspirant du « baluchonnage » québécois : la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC, prévoit l'expérimentation de prestations de « relayage » de l'aidant à domicile jusqu'à six jours consécutifs pour les situations où l'accueil temporaire en établissement n'est pas adapté à la personne aidée. Néanmoins, le Gouvernement partage avec vous, madame Guidez, le sentiment que ce que nous avons pu faire jusqu'à présent n'est pas encore suffisant. Il est temps d'agir et d'aller plus loin. Ensuite, devant un sujet aussi important et aussi complexe- car il s'agit de répondre à des situations très variées, de la personne âgée qui aide un conjoint atteint de la maladie d'Alzheimer au parent d'un enfant autiste, en passant par le salarié qui suit de près des parents vieillissants le Gouvernement a choisi d'adopter une approche structurée et, surtout, globale du sujet. Jusqu'à présent, nous avons ajouté par-ci par-là des dispositions en faveur des aidants, défini une démarche globale, sans tenir un discours global, donc sans entraîner une mobilisation globale de la société sur le sujet. Les aidants eux-mêmes ne connaissent pas bien les dispositifs et ne les utilisent pas.

Il convient désormais d'envisager le sujet dans toutes ses dimensions. Cette approche globale, associant tous les partenaires concernés, prévaut aujourd'hui dans le cadre de la concertation nationale « grand âge et autonomie », dont le pilotage a été confié à M. Dominique Libault par le Premier ministre et qui a été lancée le 1 octobre par Mme Buzyn. Cette concertation traite d'abord des personnes aidées, parce que nous pensons que la première priorité pour aider les aidants, c'est aussi d'offrir le meilleur accompagnement possible aux personnes aidées. Le Gouvernement a d'ailleurs engagé la même démarche concernant les personnes en situation de handicap : c'est l'objet du mouvement de transformation de l'offre d'accompagnement des personnes handicapées pour offrir des solutions adaptées aux besoins et aux projets de vie des personnes et de leurs proches ou des travaux engagés sur les solutions de répit, avec la mobilisation de crédits au titre de la Stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement. c'est aussi l'objet de tous les travaux engagés sur la simplification des démarches, s'appuyant sur le rapport du député Adrien Taquet et de Jean-François Serres, membre du Conseil économique, social et environnemental, Trop souvent, les aidants nous disent qu'ils sont là pour aider leurs proches, mais que le temps consacré à ceux-ci ne doit pas être uniquement du temps administratif passé en démarches, en formalités. Ce matin, lors du comité interministériel du handicap, des annonces ont été faites en la matière. pense, par exemple, à la possibilité d'attribuer des droits sans limitation de durée aux personnes ayant un handicap non susceptible d'évoluer positivement. Ces actions conduites par le Gouvernement en faveur des personnes âgées, handicapées ou malades auront assurément des effets positifs, y compris pour les aidants. Mais, au travers de la concertation « grand âge et autonomie », nous avons aussi souhaité affirmer la nécessité de traiter l'ensemble des enjeux et des problématiques concernant les proches aidants, pour apporter des réponses efficaces, cohérentes et construites avec les aidants, pour les aidants. Ainsi, au-delà de la grande consultation publique en ligne, dix ateliers thématiques ont été constitués, dont l'un porte spécifiquement sur les aidants, la famille et le bénévolat. Cet atelier réunit l'ensemble des acteurs concernés : des représentants des aidants, des associations, des acteurs locaux ou de terrain, comme les agences régionales de santé, les ARS, des conseillers départementaux, des administrations, sans oublier, bien évidemment, les parlementaires. À ce titre, le Gouvernement a souhaité confier la coprésidence de l'atelier à Mme la députée Annie Vidal. Conscient de l'intérêt porté par les parlementaires au sujet, le Gouvernement a souhaité que d'autres parlementaires puissent participer aux travaux de cet atelier en tant que membres permanents. Concernant l'atelier relatif aux proches aidants, M. le député Pierre Dharréville participera aux travaux du groupe pour l'Assemblée nationale. Le Gouvernement avait souhaité que le Sénat participe également à la concertation « grand âge et autonomie », mais, malheureusement, à ce jour, cette demande n'a pas reçu de réponse favorable, ce que nous ne pouvons que regretter. Sur le fond, l'atelier abordera l'ensemble des problématiques intéressant les aidants : il concernera tous les profils d'aidants- jeunes, salariés, non-salariés, aidants d'une personne handicapée, âgée ou malade. Il devra répondre à tous leurs besoins, à chaque étape de leur parcours, depuis l'information sur leurs droits et ceux des personnes aidées jusqu'aux solutions de répit, en incluant la question de la conciliation entre la vie professionnelle et l'aide apportée. Cette concertation doit conduire à la préparation d'un projet de loi, qui sera déposé au Parlement d'ici à la fin de l'année 2019, comme s'y est engagé le Président de la République dans son discours devant le Congrès, le 9 juillet dernier. Dans ce projet de loi, nous pourrons introduire, avec une vision globale du sujet, des mesures pour les aidants, en parfaite cohérence et en articulation avec les mesures pour les personnes aidées qui seront issues de la concertation. C'est pourquoi le Gouvernement, malgré le grand intérêt qu'il porte à ce sujet et la qualité du travail que vous avez accompli, ne peut soutenir aujourd'hui la présente proposition de loi. N'importe quoi ! Ce texte aborde des sujets importants et présente des pistes de travail intéressantes,

Surtout, comme je l'ai déjà dit, il risque d'être en décalage avec les propositions issues de la concertation « grand âge et autonomie » ou les travaux en cours sur la réforme des retraites.

L'article 1 instaure une négociation collective obligatoire régulière au niveau de la branche sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants. Le Gouvernement soutient le dispositif proposé. Aujourd'hui,

avec leur activité professionnelle. Or toutes les enquêtes le démontrent : être aidant peut emporter de nombreuses conséquences négatives sur la santé, la vie sociale, mais aussi la vie privée et la vie professionnelle. Stress, fatigue physique et/ou morale, surmenage : les salariés aidants sont davantage exposés que les autres aux arrêts maladie, mais aussi aux renoncements professionnels, à la réduction ou à la cessation totale

Il s'agit donc d'une question de responsabilité sociale et sociétale qui prend et prendra de plus en plus d'importance. Nous devons sensibiliser nos entreprises et les accompagner dans une démarche constructive, qui permette d'apporter des solutions adaptées aux besoins de leurs salariés proches aidants, et ce dans l'intérêt de tous, employés comme employeurs. L'article 1, tel que modifié par la commission, reprend désormais le cadre de l'article 33 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, censuré par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif. En soumettant expressément et spécifiquement la question de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés aidants à la négociation obligatoire régulière de branche, il donne une visibilité sans équivoque à cette question et va dans le bon sens. L'article 2 prévoit à la fois un assouplissement des conditions du congé de proche aidant, auquel je suis favorable, et une indemnisation de celui-ci par un fonds spécifique, financé par une surprime assise sur certains contrats d'assurance, mesure sur laquelle le Gouvernement est plus réservé. pas sur le principe de l'indemnisation, bien sûr, mais sur ses modalités. Créé par la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, le dispositif du congé de proche aidant a permis de soutenir la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle pour des millions de proches aidants qui travaillent. Néanmoins, ce congé est, dans les faits, très peu sollicité, et la raison le plus souvent invoquée pour expliquer ce faible recours est l'absence de compensation financière. C'est pourquoi la création d'une indemnisation du congé de proche aidant est régulièrement évoquée afin de rendre plus effectif ce dispositif. Il s'agit d'une demande forte des aidants. C'est aussi une recommandation formulée par le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, le HCFEA, dans son rapport du 12 décembre 2017 sur la prise en charge des personnes en perte d'autonomie ou, plus récemment, par Mme Dominique Gillot, dans son rapport du 19 juin dernier. Je ne peux que partager l'objectif de créer de meilleures conditions pour permettre aux aidants qui travaillent de s'occuper de leurs proches sans que cela porte préjudice à leur carrière ou à leur situation financière. Je pense d'ailleurs que le congé de proche aidant n'est pas la seule solution à privilégier et que les entreprises doivent mieux prendre en compte la situation de leurs salariés aidants. Certaines le font déjà par des aménagements d'horaires, des appuis psychologiques ou administratifs.

proposer des solutions globales. Je l'ai dit initialement, le Gouvernement préfère adopter un paquet de mesures législatives après cette concertation. Par ailleurs, les modalités de financement que vous proposez soulèvent de nombreuses interrogations. Le texte prévoit une taxe de 1,7 % assise sur certains contrats d'assurance. Il s'agit d'une piste de financement nouvelle, qui vise à préserver les finances publiques, mais elle appelle plusieurs observations. Tout d'abord, si le congé de proche aidant devait être indemnisé, la question des sources de son financement, public ou privé, devrait être discutée dans la perspective plus globale des travaux sur le financement de la dépendance menés dans le cadre la concertation. La prise en charge de nos aînés en perte d'autonomie et l'accompagnement, y compris financier, des proches aidants constituent un enjeu de société : il s'agit de faire la part entre la solidarité familiale et la solidarité nationale. Cela doit faire l'objet d'un débat national d'ampleur. Il faut mettre sur la table l'ensemble des options possibles, évaluer les dépenses prioritaires et les ressources disponibles, avant d'aboutir à la solution la plus pertinente et soutenable sur le long terme. La taxe de 1,7 % assise sur certains contrats d'assurance permettrait certainement de garantir des recettes dynamiques, à hauteur de près de 300 millions d'euros par an, selon l'exposé des motifs

cours des négociations avec les assureurs, à ce qu'il n'y ait aucune augmentation des tarifs des contrats d'assurance complémentaire santé. Le Gouvernement reste attaché à ce principe, et le dispositif proposé présente un risque fort en la matière.

Cependant, vous le savez, le Gouvernement a confié à Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites, la préparation de la mise en place d'un nouveau système universel de retraite, la coordination des travaux et la concertation avec les principaux acteurs concernés. Le Sénat a été associé à ces travaux, qui doivent aboutir à la présentation d'un projet de loi en 2019. Lors du colloque sur l'avenir des retraites organisé ici même le 19 avril dernier, immédiatement après le lancement officiel de la mission, M. Delevoye vous a indiqué les objectifs, le calendrier et la méthode de concertation et de travail retenus. les sénateurs Jean-Marie Vanlerenberghe et René-Paul Savary se sont rendus avec M. Delevoye dans trois pays européens pour observer les « conditions de réussite » des réformes engagées dans les années quatre-vingt-dix. Enfin, hier matin, la commission des affaires sociales a auditionné M. le haut-commissaire. Une deuxième phase de concertation avec les partenaires sociaux s'est ouverte le 22 octobre dernier. Son calendrier prévoit explicitement des discussions sur les nouvelles solidarités aujourd'hui nécessaires, en particulier à l'égard des aidants. Dans ce contexte, le Gouvernement considère qu'il est prématuré de modifier les règles en matière de retraites, même si nous devons garder en tête la prise en compte de la question des aidants et adopter une approche harmonisée de leur traitement, indépendamment du profil de la personne aidée.

L'article 5 ouvre aux agents publics civils l'expérimentation, prévue à l'article 53 de la loi ESSOC, de la dérogation au droit du travail dans le cadre de prestations de « relayage ». J'y suis favorable, mais il ne me semble pas nécessaire d'en passer par la loi. L'expérimentation du « relayage », inspirée de l'exemple du « baluchonnage » québécois, a en effet été mise en place par la loi ESSOC, adoptée le 10 août 2018. Il s'agit de répondre au besoin de relayer les aidants dont la charge est la plus lourde, en raison du besoin de présence ou de soins constants à leur domicile requis par la situation de la personne aidée. L'article 53 de cette loi permet à titre expérimental, dans plusieurs départements volontaires qui seront déterminés après appel à candidatures, aux établissements et services d'aide de recourir à des salariés volontaires pour assurer des prestations de suppléance de l'aidant à domicile par un seul et même personnel, sur une période pouvant aller jusqu'à six jours consécutifs. Pour ce faire, il a fallu prévoir des dérogations au droit du travail, qui ne concernent pas les agents publics, puisque les règles relatives à leur temps de travail relèvent non pas du domaine législatif, mais du pouvoir réglementaire autonome. J'accueille donc avec grand intérêt votre proposition, qui permettrait d'élargir le cadre de l'expérimentation de manière harmonisée aux secteurs public et privé, mais il n'y a pas besoin de la loi pour cela. Il me paraît par ailleurs tout de même nécessaire d'avoir des échanges avec échanges avec le ministre chargé de la fonction publique, d'une part, et avec les représentants de chaque fonction publique, en particulier des fonctions publiques territoriale et hospitalière, part. L'article 6, tel que revu par la commission des affaires sociales, prévoit l'enregistrement sur la carte Vitale de la personne aidée du nom de l'aidant et/ou de la personne de confiance. Son dispositif incite à la déclaration d'une personne de confiance, automatise l'envoi d'un guide de l'aidant et préconise la mise en place d'un portail d'information et d'orientation à destination des aidants. J'ai aussi quelques réserves La question de l'identification des aidants et de leur accompagnement est importante. Il faut en effet pouvoir repérer les fragilités des aidants, prévenir les conséquences de la fatigue physique ou psychologique liée

Sur un autre point soulevé par cet article, le Gouvernement partage bien évidemment l'objectif de renforcer l'information des aidants. Des efforts ont été réalisés sur ce point. La loi du 28 décembre 2015 a consacré et renforcé le droit à l'information des personnes âgées, de leur famille

Au niveau national, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, a été chargée de développer un portail d'information,, qui comporte un volet spécifique sur l'information destinée aux aidants. Certes, ce portail ne s'adresse pas à tous les aidants. C'est pourquoi, à partir de cette expérimentation, le Gouvernement travaille à la création d'un portail national pour améliorer l'information des personnes handicapées et de leurs familles, tel qu'évoqué dans la proposition 7 du rapport du comité Action publique 2022 de juin 2018.

ont remis au printemps dernier. Nous en sommes aujourd'hui à la mise en oeuvre de ses recommandations. La simplification des parcours et des démarches, la lisibilité des dispositifs seront aussi parmi les enjeux de la concertation « grand âge et autonomie » lancée le 1 octobre

Par exemple, dès lors que l'information peut être disponible en ligne, se posent les questions de la pertinence de l'envoi systématique d'un « guide de l'aidant » et du coût Pour toutes ces raisons, et même si les questions abordées devront trouver des réponses dans le cadre des ateliers de la concertation, le Gouvernement ne peut soutenir les dispositions prévues par cet article.

Dans ce contexte, le Gouvernement ne peut pas être favorable à cette proposition de loi. Je profite de l'examen de ce texte pour réitérer, madame Guidez, l'invitation du Gouvernement à travailler ensemble, de manière constructive, à l'élaboration d'une politique globale en faveur des proches aidants dans le cadre de la concertation. enrichir les idées du Parlement ! Cela nous permettra d'aborder de nouveau le sujet lorsque la concertation aura permis d'aboutir à une stratégie complète, avec des solutions entièrement partagées, pragmatiques, efficaces et soutenables financièrement sur le long terme.

qui a eu le courage de s'attaquer à la problématique des proches aidants. Cette problématique, nous le savons tous, est un serpent de mer des politiques d'accompagnement de la dépendance, alors que 9 millions de Français accompagnent aujourd'hui un proche âgé ou dépendant- 9 % à y consacrer plus de quarante heures par semaine. Pour ceux-là et pour tous les autres, il était du devoir du Parlement de se saisir de cette question.

En se mettant au service de l'autre, ils ne peuvent plus subvenir aux besoins de leur foyer. Sans statut, sans revenu, simplement sans droits, ils ne peuvent pas trouver leur place dans le dispositif actuel d'accompagnement. La création d'une indemnité associée au congé de proche aidant est donc une étape essentielle pour reconnaître leur contribution au bon fonctionnement de notre société. Différentes étapes ont jalonné ce parcours vers la reconnaissance des proches aidants.

Un décret du 9 octobre dernier a encore amélioré cette situation, en ouvrant le dispositif de don de jours de congé aux fonctionnaires. Aujourd'hui, il est temps de franchir une nouvelle étape, en instaurant une indemnité pour le proche aidant. Cette proposition de loi répond à un impératif de société. le nombre d'aidants en charge de l'accompagnement d'un proche âgé ou dépendant est, cette année encore, en hausse de huit points, et cette charge devient de plus en plus lourde pour les proches : 31 % des aidants familiaux reconnaissent ainsi négliger leur santé, être victimes de stress, de manque de sommeil ou de douleurs physiques. Si l'État providence doit être repensé, la protection des publics fragiles doit rester sa mission sacrée. Nous ne devons jamais les abandonner ! Pour être à la hauteur du dévouement de ces proches aidants, les auteurs de la proposition de loi souhaitent C'est une mesure essentielle, et la commission des affaires sociales a su compléter intelligemment ce dispositif. L'ensemble des amendements proposés par le rapporteur a ainsi été adopté, afin de simplifier les mécanismes de financement de l'indemnité, de définir la surcote en taxe et de fixer son taux, mais aussi d'éclairer la situation de fin anticipée de congé d'un proche aidant. Pour, demain, mettre en oeuvre ce nouveau modèle de financement de l'accompagnement, il faudra surveiller la trajectoire financière de ce dispositif, la pérennité est la clé de voûte de la fonctionnalité. La proposition de loi y pourvoit, en majorant la durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Voilà donc une proposition humaine et sociale, à l'écoute des réalités de terrain, financièrement gagée et fiscalement équilibrée pour préserver l'équilibre des comptes publics. Cet édifice ne serait pas complet sans un volet informatif. Là encore, la proposition de

Ce rôle, assumé par les membres de la famille ou par des proches, est à la fois indispensable et éreintant. Comment concilier la vie professionnelle et le quotidien d'aidant ? Comment ne pas céder à l'oubli de soi ? Comment assurer une présence affective lorsque la fatigue arrive, lorsque le sentiment d'« insolitude » se fait sentir, lorsqu'aucun répit n'est finalement autorisé et que la culpabilité s'immisce peu à peu, lorsqu'aucun soutien ou aucun relais n'est envisageable Cette situation appelle une réaction, demandée de longue date par les associations d'aidants. Je tiens donc à saluer le formidable travail réalisé par nos collègues Jocelyne Guidez et Olivier Henno. Au regard de la pyramide des âges, nous constatons que les baby-boomers aidants de ces deux dernières décennies sont les personnes dépendantes de demain. Leur fort poids démographique doit nous faire prendre conscience que la gestion de la dépendance se fera en renforçant

dans un domaine qui relève d'une évidente solidarité témoignée à un parent en situation de handicap, et cela sans attente d'un retour. Charge au législateur de trouver la juste distance pour ne pas créer un carcan, tout en accompagnant et protégeant. Les « proches donnants », si vous me permettez cette expression, souffrent de ne pas pouvoir accéder à des moments de répit, et 56 % d'entre eux admettent subir, en plus de cette détresse psychologique, une dégradation de leur situation financière. C'est pourquoi créer un dispositif d'indemnisation du proche aidant et donner à celui-ci un statut clairement identifié et identifiable est à mes yeux primordial.

À l'heure des comportements trop souvent individualistes, ne pas reconnaître leur action serait un mauvais signal. Malgré les difficultés de la tâche, épauler quelqu'un est un acte gratifiant,

fait sens avec notre époque, avec notre société si complexe au regard des âges différents qui la composent. Je vous invite, à mon tour, à adopter ce texte, qui en appelle bien d'autres pour améliorer la situation des proches aidants.

madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Jocelyne Guidez, modifiée par la commission des affaires sociales, vise l'objectif, largement partagé, d'accroître la reconnaissance et le soutien que notre société doit apporter aux proches aidants, s'agissant notamment de leurs droits sociaux. Selon les estimations et les statistiques, encore trop lacunaires ou anciennes, 8,3 millions de personnes soutiennent et accompagnent au quotidien un proche en perte d'autonomie en raison d'une maladie, d'un handicap, d'un accident ou de son âge. Les aidants sont le plus souvent des membres de la famille, des conjoints ou des amis. Les femmes sont les premières pourvoyeuses d'aide au sein de la famille : environ 57 % des aidants sont des femmes, et leur contribution est plus forte, notamment en volume horaire. Parmi ces 8,3 millions de personnes, on compterait 4 millions de personnes salariées, dans toutes les catégories socioprofessionnelles. Or, nous le savons, les risques de ruptures professionnelles et d'isolement sont particulièrement importants pour les proches aidants.

pour offrir un répit aux aidants. Ces propositions sont le fruit de l'engagement de notre collègue Jocelyne Guidez, dont je tiens à saluer le travail sur cet enjeu social et sociétal majeur. Si nous partageons l'objectif d'améliorer au plus vite l'aide financière, matérielle et sociale des aidants, notre groupe émet des réserves sur l'adoption de cette proposition de loi, qui, à notre avis, comporte un risque de fragmentation supplémentaire de la question des proches aidants. En effet, la reconnaissance progressive du rôle des aidants a conduit à l'adoption de mesures législatives dispersées et cloisonnées, qu'il s'agisse de projets de loi ou de propositions de loi, comme celle que nous avons récemment adoptée sur le don de jours de congé. Nous sommes d'avis que cette technique des petits pas a atteint à la fois son objectif et sa limite : le sujet des aidants est désormais incontournable

Ce plan global, annoncé par le Gouvernement, devra également actualiser et harmoniser le cadre juridique applicable et améliorer la gouvernance et la cohérence des politiques publiques d'aide aux aidants. Sur le terrain, en effet, les aidants ont ont cruellement besoin d'un interlocuteur unique pour s'y retrouver dans le maquis des acteurs publics et privés du handicap et de la dépendance. J'ajoute que le sujet des aidants est indissociable de celui des politiques publiques en matière de perte d'autonomie et de handicap. Là encore, un chantier majeur est en cours, et la question des aidants ne peut être traitée indépendamment de lui. Comme l'a souligné le Haut Conseil de la famille, « le premier droit des aidants est que le plan d'aide de leur proche soit d'un bon niveau et qu'un service public de bonne qualité le mette en oeuvre ». Je partage l'avis émis par notre collègue député Pierre Dharréville dans son rapport de « mission flash » sur les aidants : « Les personnes aidantes fournissent un travail gratuit, un travail informel qui vient au mieux en complément, au pire en palliatif d'une réponse publique qui n'est pas à la hauteur ». Eh oui ! On ne peut durablement faire reposer une part significative de la prise en charge de la perte d'autonomie sur les épaules des personnes aidantes. Je le répète : si l'action publique doit, bien entendu, venir en aide aux aidants, ce ne peut être sa fin ultime

d'une « mission flash » pilotée par Pierre Dharréville, suivie d'une proposition de loi. Ces deux initiatives de l'Assemblée nationale ont permis d'identifier les difficultés rencontrées par les proches aidants et de proposer des solutions. Le constat fait à l'époque est que les proches aidants pallient bien souvent les carences des professionnels de santé et des institutions, en gérant les problématiques liées à la dépendance, dont la responsabilité incombe pourtant à l'État. Parce que les proches aidants assument un si grand rôle, il est nécessaire de leur assurer des conditions d'existence dignes, pour le présent, mais aussi pour le futur. Afin d'arriver à cet objectif, trois axes de travail ont été dégagés dans le cadre de la « mission flash » : le temps du proche aidant et son droit au répit ; les ressources dont il dispose pendant son congé et ses droits à retraite ; enfin, son encadrement, sa reconnaissance auprès des professionnels de santé et sa réinsertion dans le monde du travail, une fois sa tâche accomplie.

Nous nous félicitons de ces avancées, mais regrettons que cette proposition de loi ne tienne pas compte de l'ensemble des solutions avancées par la « mission flash ». Ainsi, il conviendrait d'assouplir les conditions de mise en oeuvre du congé, afin de faciliter son articulation avec le temps de travail. que certains aidants ont besoin d'utiliser leur congé de manière très fractionnée, à hauteur d'un ou de deux jours par semaine, le recours fractionné au congé est conditionné à l'accord de l'employeur. ailleurs, au-delà d'un « relayage » permettant aux aidants de se reposer, les frais relatifs à leur santé physique et mentale devraient être pris en charge à 100 %, afin d'éviter que leur investissement auprès de leurs proches ne les fragilise. Enfin, la reconnaissance de la lourde tâche assumée par les proches aidants passe non pas seulement par la majoration de leurs droits à retraite, mais aussi par la mise en place de dispositifs permettant leur réinsertion dans l'emploi après un arrêt prolongé et la reconnaissance des compétences acquises au cours de cette expérience. Même si nous regrettons que certains aspects de la situation des proches aidants aient ainsi été laissés de côté, cette proposition de loi constitue pour eux une avancée considérable. Certes, elle ne Certes, elle ne va pas assez loin selon nous, mais elle est créatrice de droits réels et nouveaux. C'est un premier pas. La création de droits nouveaux pour les citoyens étant une préoccupation majeure de notre groupe, il nous paraît nécessaire de soutenir toute proposition en ce sens, indépendamment de toute considération dogmatique !

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, d'après le baromètre 2017 des aidants réalisé par la Fondation APRIL, le phénomène de l'« aidance » toucherait près de 11 millions de Françaises et de Français.

Les aidants représentent une véritable alternative solidaire spontanée face aux carences de notre système d'accompagnement des personnes dépendantes. Le service gratuit rendu par ces personnes est gigantesque pour la société : si l'État devait prendre à sa charge l'accompagnement assuré par les aidants, il y consacrerait plusieurs dizaines de milliards d'euros À l'heure des restrictions budgétaires, aider les aidants se révèle donc autant une mesure d'épargne publique que de salut public. C'est d'autant plus vrai que, par ailleurs, les projections démographiques confirment que ce phénomène sociétal va s'amplifier, du fait de l'augmentation exponentielle des maladies chroniques et du vieillissement de la population. D'ici à 2060, le nombre de personnes en perte d'autonomie devrait doubler, pour dépasser les 2,5 millions. Il faut donc saisir à bras-le-corps ce sujet d'avenir, au plus vite ! Cette proposition de loi vous y invite, madame la secrétaire

initiative d'ailleurs repoussée par le Gouvernement dans l'attente d'un projet de loi sur le cinquième risque « perte d'autonomie », dont on attend toujours la première mouture ... Alors qu'une concertation est lancée sur le thème du grand âge et de l'autonomie, le Sénat se donne l'occasion d'apporter sa contribution. Il s'agit également d'inciter le Gouvernement à accélérer ses réflexions, en vue de proposer des solutions concrètes aux aidants, et à se prononcer sur les mesures dont nous aurons à débattre dans quelques instants. Le législateur n'est pas resté inactif ces dernières années sur la question. Dès 2015, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement a consacré la définition juridique des aidants et transformé le congé de soutien familial en congé de proche aidant. le don de jours de repos à un collègue a été étendu aux proches aidants par la loi du 13 février 2018. Mais est-ce bien suffisant ? Nous pensons que non, et que l'on peut toujours mieux faire. Il faut désormais aller plus loin, et, une fois n'est pas coutume, la Commission européenne nous y invite, avec la publication, en avril 2017, du socle européen des droits sociaux, qui comprend un volet spécifique sur les aidants. La prise de conscience est donc bel et bien générale et transpartisane. Cette proposition de loi participe de cette volonté de répondre à l'urgence sociale. Il ne s'agit pas d'entretenir une vision doloriste de l'aidance, mais de reconnaître pleinement les aidants dans leur solidarité, de faciliter leur quotidien

ailleurs, l'extension de la durée du congé, l'assouplissement des modalités de recours, l'intégration de la conciliation des vies personnelle et professionnelle des aidants dans la négociation collective, la meilleure information et la validation de périodes d'assurance pour le calcul des droits à pension sont autant de droits nouveaux essentiels qui faciliteront grandement la vie de l'aidant. La situation des aidants, qui est souvent vectrice d'inégalités, suscite des conséquences dans leurs vies personnelle, professionnelle et sociale. Toujours sollicité, parfois même accaparé, le proche aidant s'oublie lui-même et relègue au second plan sa santé, mais surtout sa vie.

La reconnaissance de l'aidant doit permettre à la société dans son ensemble, et au monde de l'entreprise en particulier, de changer de regard sur l'aidance. Les compétences déployées par les aidants en matière d'organisation, d'arbitrage et de décision doivent être valorisées.

dans ce domaine, afin de rendre non pas hommage, mais justice à ces piliers invisibles et néanmoins indispensables de la solidarité nationale

qui s'inscrit dans le prolongement du rapport qu'elle a présenté il y a neuf mois sur la proposition de loi de Paul Christophe ouvrant le don de jours de congé payés entre salariés au bénéfice des proches aidants. M'exprimant à cette tribune lors de la discussion générale, j'avais alors estimé que cette proposition de loi allait dans le bon sens, tout en reconnaissant qu'elle laissait en suspens un certain nombre de questions, auxquelles votre texte, ma chère collègue, tente de répondre. Vous proposez notamment que la question des aidants soit intégrée au champ obligatoire des négociations collectives- c'est l'article 1 du texte -et que le congé de proche aidant soit indemnisé- c'est son article 2 -, permettant ainsi d'améliorer la situation de ces personnes plus que jamais indispensables au bien-être Les proches aidants jouent un rôle fondamental, que l'État ne peut entièrement assumer, d'autant moins que, avec le vieillissement de la population, leur nombre est amené à s'accroître dans les années à venir. Il est donc nécessaire de donner sans plus attendre davantage de moyens aux proches aidants pour assumer leur rôle. Toutefois, il ne s'agit pas uniquement de leur faciliter la tâche. En effet, ces aidants, encore souvent en activité, éprouvent des difficultés à concilier travail et obligations familiales.

22 % déclarent avoir été obligés de reporter des soins qui les concernaient ; 11 % font état de problèmes de santé survenus depuis qu'ils sont aidants. L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé a même évoqué un risque de surmortalité des aidants par rapport à la population générale ainsi, un tiers des aidants décéderaient avant la personne qu'ils soutiennent. C'est pourquoi il est essentiel que les aidants soient à leur tour soutenus, aidés, accompagnés et mieux informés. proposition de loi prévoit la mise en place d'un guide de l'aidant et d'un site internet d'information et d'orientation. C'est très bien, compte tenu de la forte demande des aidants, qui se sentent souvent démunis. démunis. Ce nouveau texte n'est pas sans rappeler la proposition de loi du député Pierre Dharréville en faveur d'une reconnaissance sociale des aidants, examinée à l'Assemblée nationale le 8 mars dernier,

Je ne puis souscrire à cet argument : comme je l'ai dit en commission, le législateur ne peut se contenter d'attendre les initiatives du Gouvernement ! En outre,

Comme l'a justement expliqué notre rapporteur, « ce texte suggère que nous embrassions d'un seul regard une palette de droits nouveaux pour tous les aidants, leur offrant ainsi le seul vecteur possible de progrès

problème s'ajoute la question, centrale pour nous, du vieillissement en terre d'immigration : de nombreux immigrés qui se sont installés sur mon territoire vont y finir leur vie,

de faciliter l'hébergement temporaire en EHPAD et de favoriser le remplacement des aidants familiaux par des professionnels pendant quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. Bien des choses restent à accomplir pour valoriser les emplois d'aide à domicile et pour mieux informer sur les aides disponibles. Parce à la solitude, à l'épuisement des aidants familiaux, et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, je n'ai pas hésité une seule seconde à cosigner ce texte. Madame la secrétaire d'État, nous pouvons évidemment comprendre les contraintes de calendrier du Gouvernement, mais le législateur se doit d'être aussi force de proposition.

Cela sera malheureusement de plus en plus le cas, compte tenu du vieillissement de la population et de l'augmentation des maladies chroniques et neurodégénératives. S'appuyer sur des proches aidants sera une nécessité croissante. Selon une étude, le travail des aidants familiaux représente entre 0,6 % et 0,8 % de notre PIB. Il s'agit d'un travail non reconnu, dont la valeur atteint chaque année entre 12 et 16 milliards d'euros. Citer ces chiffres, alors que chaque histoire est unique et personnelle, donner une valeur monétaire à ces actes, alors qu'ils sont des preuves d'amour et de solidarité, me trouble et m'interpelle. À travers la singularité des parcours, ces chiffres jettent un regard froid et direct sur l'universalité de la condition humaine. Je salue donc tout particulièrement l'engagement de notre collègue Jocelyne Guidez, qui, depuis le début de son mandat, début de son mandat, a travaillé sans relâche sur cette problématique. Au moment où nous mettons en place une nouvelle stratégie de santé, plus tournée vers la prévention, cette proposition de loi est une main tendue pour répondre à un enjeu social et sociétal majeur. Il s'agit de favoriser la reconnaissance des proches aidants, de les épauler dans leur mission et de leur apporter le soutien qui leur est dû. Il s'agit, mes chers collègues, madame la secrétaire d'État, d'être à la hauteur de la situation.

je tente de la raconter, mais chacun d'entre vous pourrait le faire. L'aidant est une personne naturellement désignée qui accompagne un proche fragilisé. Bien souvent, il ne se rend pas compte qu'il est un aidant, il est le parent, le conjoint, l'enfant, l'ami, le voisin. Ce proche endossera la responsabilité des démarches administratives de l'aidé au moment où le récent diagnostic affectera profondément Il s'occupera des courses, du lever, du coucher, du repas, de la toilette et, souvent, il s'oubliera lui-même, remettant à plus tard ses propres rendez-vous médicaux, ses loisirs, sa vie, en somme. Le risque d'isolement et de traumatisme psychologique est important.

Si je quitte mon emploi, de ma retraite ? Qui peut m'aider ? Dans ces péripéties de la vie, le proche aidant forme un duo avec l'aidé, mais seul ce dernier est visible, reconnu et pris en charge. Est-ce juste ? Non. Aussi, en

qui distinguent et référencent les initiatives positives. Les collectivités s'organisent aussi en s'appuyant sur des fondations ; des conseils départementaux à la conférence des financeurs, beaucoup d'initiatives se font jour, sur tous les territoires. Des groupes de parole et des temps forts sont mis en place, mais cela n'est pas suffisant. Les proches aidants sont au coeur de cette proposition de loi. Notre rapporteur, Olivier Henno, a détaillé le dispositif dont je rappellerai seulement les objectifs : détecter l'aidant le plus rapidement possible ; lui fournir les éléments nécessaires pour qu'il puisse se faire accompagner, ainsi qu'un soutien financier pour qu'il ne mette pas son propre avenir en péril ; lui permettre d'être reconnu sans crainte dans son entreprise et auprès des médecins de l'aidé

Ce qui se joue aujourd'hui, c'est non pas l'adoption d'un texte par un Sénat d'opposition, mais l'adoption d'un texte par des représentants de la République, unis autour d'une cause commune. Nous devons prendre une décision pour que, à l'avenir, notre société soit juste et humaine, humainement juste et justement humaine.

8,3 millions de nos concitoyens répondent à la définition de « proches aidants », en ce qu'ils apportent une aide humaine sans pour autant en tirer un salaire. Cette définition date de la loi du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement. En janvier dernier, nous ajoutions une pierre à l'édifice du statut des proches aidants en adoptant la proposition de loi déposée par notre collègue Paul Christophe, dont l'objet était de créer un dispositif de don de jours de repos non pris, à leur bénéfice. La proposition

Notre collègue Jocelyne Guidez, auteur de la proposition de loi, que j'ai d'ailleurs cosignée, s'est attelée à un travail minutieux et précis, en réponse aux attentes légitimes des proches aidants. Je salue sa détermination et les mécanismes innovants qu'elle nous soumet sur ce sujet important. Elle a été secondée dans sa démarche par notre rapporteur Olivier Henno, que je félicite de son travail rigoureux. Le rôle des proches aidants est essentiel, en ce qu'ils viennent suppléer les manquements de nos politiques sociales dans le domaine du vieillissement, du handicap ou de la maladie. eux se retrouvent dans des situations difficiles financièrement, parce qu'ils ont été contraints de cesser toute activité professionnelle, moralement, parce qu'ils consacrent tout leur temps à la personne aidée, et physiquement, parce qu'ils ne peuvent pas souffler ou qu'ils ne connaissent pas les gestes professionnels à effectuer. Le temps qui m'est imparti ne me permet pas d'aborder l'ensemble des articles de ce texte ; j'insisterai donc sur deux points spécifiques. Tout d'abord, la principale avancée de cette proposition de loi réside selon moi dans l'instauration d'une indemnisation du congé de proche aidant, à l'article 2. Le financement de cette indemnité est assuré et innovant : il repose sur un droit de tirage de l'employeur sur un fonds spécifique alimenté par une surcote portée à un niveau maximum de 1,7 % sur les primes de produits assurantiels. Ainsi, les finances de l'État ne sont pas sollicitées. Je retiendrai ensuite l'article 4, qui prévoit les modalités d'uniformisation d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de tous les proches aidants, quelle que soit la personne qu'ils accompagnent et leur statut professionnel. Cet article met fin à une discrimination au regard de la retraite entre les proches aidants de personnes en perte d'autonomie et ceux de personnes handicapées. Je salue cette avancée.

à nous proposer un texte dans les mois qui viennent, en espérant que celui-ci soit à la hauteur des enjeux que nous avons évoqués aujourd'hui. Au regard de cette situation, pour affirmer son positionnement et l'intérêt qu'il porte à cette proposition de loi, le groupe Les Républicains

qu'il existe un droit constitutionnel du Parlement, qui a été mis en place par un président dont on disait qu'il n'était pas un grand démocrate, à savoir Nicolas Sarkozy.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le 31 janvier dernier, à l'occasion de la discussion de la proposition de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap, je confirmais l'importance du sujet des aidants familiaux et la nécessaire évolution législative de leur statut, au regard de leur importance croissante pour nos populations et nos territoires. j'ai d'ailleurs remarqué que toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi avaient été prises par le Gouvernement. Il ne manque que la publication du rapport visant à évaluer la possibilité de réviser l'imposition des sommes versées à titre de dédommagement dans le cadre de la prestation de compensation, afin de soutenir et de valoriser les proches aidants. J'ose espérer, madame la secrétaire d'État, que, eu égard au sujet, ledit rapport paraîtra bientôt. Je ne suis pas non plus convaincu, à titre personnel, que le développement des maisons de retraite et des EHPAD soit le symbole d'une évolution positive de notre société. Bien au contraire, je considère que l'avenir du bien-être de nos populations âgées réside dans la création d'un réel statut de l'aidant, ainsi que dans la mise en oeuvre de mécanismes de protection

que le vieillissement de la population française s'intensifie, notamment aux Antilles, lesquelles se classent parmi les régions les plus âgées de France. En 2014, quelque 92 180 personnes âgées de soixante ans et plus résidaient en Martinique,

Mme Jocelyne Guidez. Cet amendement tend à insérer la possibilité de rendre prioritaires au compte personnel de formation- ou CPF -les salariés qui se seraient absentés au titre des congés sociaux non rémunérés. Il vise clairement les proches aidants, issus aussi bien du secteur privé que du secteur De nombreux aidants actifs que j'ai rencontrés m'ont sollicité à ce sujet. Nous leur devons ce droit de priorité, en raison de leur investissement au quotidien auprès de leur proche, pour qu'ils ne perdent pas pied dans le monde du travail, et, enfin, parce que cette évolution est attendue et souhaitée. Il s'agit non pas de créer des inégalités entre salariés, mais bien de permettre à ceux qui se sont absentés pour des raisons éminemment humaines, de bénéficier d'abord de ces formations, afin de se remettre à niveau. Une absence d'un an, de deux ans, de trois ans- parfois plus encore les techniques professionnelles évoluent vite. J'ai récemment participé à une rencontre dans mon département de l'Essonne avec des salariés et des employeurs sur le thème de la place des proches aidants dans l'entreprise. Les témoignages étaient saisissants et bouleversants, et j'ai été agréablement surprise de voir ces chefs d'entreprise soutenir cette proposition. Ce sujet suscite une véritable attente, et il est temps de combler notre retard. Les droits sociaux doivent prendre en compte ces besoins

Conformément au principe de solidarité gouvernementale, comme vous l'avez précisé, vous soutenez l'objectif de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. J'attends donc l'expression d'un avis favorable du Gouvernement sur l'article 1. Quel

Sans indemnisation, les proches aidants ne déclenchent pas ce congé ; pis, ils sont susceptibles de recourir à des congés maladie de complaisance. Aussi, madame la secrétaire d'État, à la suite de votre intervention, je prends acte de votre soutien à l'évolution des conditions du congé de proche aidant. Je note surtout l'engagement que vous venez de prendre s'agissant de son indemnisation. Toutefois, je regrette qu'il ne s'agisse que de paroles et non d'amendements du Gouvernement

Mme Nadine Grelet-Certenais. Cet amendement vise à rétablir le texte initial de la proposition de loi, en offrant la possibilité au proche aidant de cumuler l'indemnité perçue au titre du congé de proche aidant avec la prestation de compensation du handicap, ou PCH, ou la rémunération versée au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, de la personne aidée. Parler d'effet d'aubaine pour les aidants me paraît assez inapproprié. Soutenir les aidants est un enjeu d'intérêt général, mais aussi intime. On le sait, être aidant n'est pas un choix, c'est d'abord une situation subie. C'est la raison pour laquelle il faut permettre à l'aidant de faire face à la perte d'autonomie de la personne aidée. Nous savons quel investissement personnel représente cette tâche. Nous connaissons le chiffrage en milliards d'euros des services accomplis par les aidants et l'importance du taux de non-recours aux aides. Il nous semble juste de permettre aux aidants d'obtenir une prestation prestation compensatoire et de sauvegarder le droit à la PCH ou à l'APA du parent aidé et, ainsi, de faciliter la vie de ceux qui doivent accompagner leurs proches. On peut enfin considérer que le terme de « cumul » est totalement inapproprié, car les prestations ne s'adressent pas du tout aux mêmes bénéficiaires.

Guillaume Arnell. L'article 2 met en place un fonds spécifique pour financer le congé de proche aidant. Il est prévu que ce fonds soit administré par un conseil de gestion composé à parité de représentants de l'État et de représentants d'employeurs et de salariés. Cet amendement vise à y associer les usagers. l'avis de la commission ? Cet amendement tend à associer les associations représentatives d'usagers à la gestion du fonds spécifiquement dédiée au financement de l'indemnité de proche aidant.

Mme Nadine Grelet-Certenais. Cet amendement vise à rétablir la suppression du nombre de renouvellements possibles du congé de proche aidant du champ de la négociation collective, ouvrant ainsi la possibilité d'un nombre de renouvellements non plafonnés dans la limite de trois années. Les besoins étant compliqués à évaluer et à planifier, ne pas plafonner le nombre de renouvellements possibles sur une durée de trois années permettrait au proche aidant de bénéficier de souplesse dans l'organisation de son emploi du temps professionnel et, ainsi, d'une certaine réactivité face aux aléas de santé de l'aidé. Déterminer le nombre de renouvellements possibles revient à exiger du proche aidant la capacité d'anticiper sur les périodes de dépendance plus aiguës, d'autant plus qu'une personne ayant assumé la charge d'aidant est souvent amenée à être sollicité une nouvelle fois par la famille ou par les proches. Il faut également évoquer le cas du cumul des personnes aidées, par exemple un enfant et une personne âgée. La suppression du nombre de renouvellements possibles du congé de proche aidant du champ de la négociation collective offre une réelle flexibilité et permet, à terme, l'instauration d'un climat plus solidaire et plus propice à l'épanouissement du proche aidant dans l'entreprise. Par conséquent, restreindre le champ de la négociation collective ouvre le champ de l'apaisement individuel, sans porter préjudice à l'équilibre existant au sein de l'entreprise. Retirer cette charge morale au proche aidant augmentera sa disposition à travailler, la sérénité étant la clé de voûte de sa bonne santé physique, d'une part, et psychologique, d'autre part.

afin de ne pas ouvrir pour la branche la possibilité de renouveler ce congé à l'infini. Cette rédaction non seulement permet une meilleure prévisibilité de la mesure pour les employeurs, mais écarte le risque

Ce programme prévoit la mise en place d'une politique d'accompagnement professionnel spécifique des jeunes sortis du système scolaire et des personnes à la recherche d'un emploi. L'objectif est de mettre au coeur des politiques publiques de l'emploi la problématique de l'aidance. Nous l'avons déjà évoqué il y a quelques instants, la prévention évite l'exclusion, au même titre que l'accompagnement favorise l'épanouissement de l'individu qui se trouve dans une situation particulièrement complexe. Faire apparaître explicitement la situation du jeune aidant ne peut que renforcer le besoin qui est le sien d'un accompagnement spécifique. Monsieur le rapporteur, La loi prévoit désormais la possibilité pour l'État de financer un programme national destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes décrocheurs ou de personnes n'ayant pas le baccalauréat. Le public cible de ce programme est défini

Toujours inspiré du rapport de Dominique Gillot, le présent amendement a pour objet de veiller à ce que les salariés qui courent un risque de désinsertion professionnelle pour cause de maladie, d'accident ou de handicap diagnostiqué, ou dont l'état de santé au travail le justifie, bénéficient d'une reconversion ou d'une promotion sociale ou professionnelle grâce à des actions de formation spécifiques. Le proche aidant exerce, d'une certaine façon, et à titre gracieux, des tâches pour lesquelles il n'est ni qualifié ni prédisposé en raison de sa vie privée et de son organisation professionnelle. Nombre de spécialistes, tels que l'interne en médecine Hélène Rossinot, constatent que le proche aidant atteint souvent un point de non-retour, en s'oubliant lui-même et en reléguant sa santé au second plan. Ces reports de soins, fréquents, entravent la détection des maladies graves. Si préserver la santé des aidants est un enjeu de santé publique aujourd'hui, leur permettre d'être maintenus à un poste qui leur correspond, ou de changer de métier ou de profession, ou encore de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle, nous la réponse la plus efficace. En effet, nous le savons : s'adapter au nouvel état de santé de l'aidant empêche sa mise à l'écart et prévient l'exclusion professionnelle. Les réflexions doivent s'orienter vers un meilleur encadrement dans le cadre de la reconversion professionnelle.

Guidez, sur l'article. Comme l'article 4, l'article 3 s'attache aux droits sociaux des aidants et, particulièrement, à leur retraite. Alors que ces dispositions ont notamment été à l'origine du renvoi en commission d'une proposition de loi en début d'année à l'Assemblée nationale,

la question des droits ultérieurs et, en particulier, celle de la retraite. On sait bien, en effet, que s'occuper d'une personne en situation d'extrême handicap nécessite du temps, ce qui se fait souvent au préjudice de la carrière professionnelle. Il n'y a pas de raison de pénaliser pénaliser l'ensemble des aidants. Il faut donc être attentif à ce que ces dispositions soient prises en compte. Comme l'évoquait à l'instant Jocelyne Guidez, il est important que, à l'orée d'une réforme des régimes de retraite,

madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, permettre à un professionnel de remplacer un aidant à domicile plusieurs jours d'affilée, afin que celui-ci puisse partir l'esprit léger et tranquille, se ressourcer, s'occuper de lui, est, à l'heure actuelle, un rêve inaccessible pour la majorité des aidants. La faute en revient à un cadre réglementaire inadapté et à un manque de financements. la réglementation en vigueur contraint actuellement à faire se succéder plusieurs relayeurs auprès d'un aidé en cas d'absence de l'aidant principal, conformément aux conventions collectives des services à la personne, qui limitent la durée maximale de présence continue à dix ou douze heures. Or, comme le soulignait la députée Joëlle Huillier dans son rapport au Premier ministre, « les relayeurs expriment tous le fait qu'ils vivent les temps de présence trop courts comme une forme de maltraitance. [ ...] Le consensus semble se faire sur un idéal d'un seul intervenant sur une durée de trente-six Dès lors, il est nécessaire que l'État, les collectivités locales et les partenaires sociaux du secteur de l'aide à domicile se coordonnent et s'engagent dans un échange constructif pour contribuer à faire évoluer cette situation. Pour ce faire, il est également nécessaire de pouvoir s'appuyer sur des travaux documentés et solides, afin d'apporter les modifications législatives nécessaires à l'encadrement du statut de relayeur. il est nécessaire d'harmoniser le coût du service de relayage, afin que le reste à charge pour les familles soit raisonnablement acceptable, grâce à un financement pérenne et régulier prévu dans le cadre d'une politique publique de subventionnement en faveur de l'aide au répit et, plus particulièrement, de l'aidant. L'expérimentation L'expérimentation prévue à cet article est nécessaire pour parvenir à une analyse plus fine et précise de l'ensemble de ces éléments, et apporter des solutions adaptées pour favoriser le développement du relayage. Je mets aux voix

Le présent amendement a pour objet de permettre à la conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées d'utiliser une partie des ressources qu'elle reçoit de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, au titre de la section V de son budget, pour financer des actions en faveur des proches aidants. Je rappelle que cette conférence des financeurs a pour objectif de coordonner, dans chaque département, les financements de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées de soixante ans et plus, autour d'une stratégie commune. Il y a donc une vraie logique à permettre une action globale, coordonnée et partagée pour les acteurs locaux. Cette faculté qui serait reconnue à la conférence départementale des financeurs pourrait faciliter le financement d'actions de prévention de l'épuisement physique ou psychique auquel sont fréquemment exposés les proches aidants. Elle s'inscrirait en parfaite complémentarité avec la mission première de la conférence des financeurs, qui vise avant tout à financer des actions de prévention de la perte d'autonomie. Une telle disposition exprimerait une forme de reconnaissance supplémentaire du rôle essentiel joué par les proches aidants, en favorisant le renforcement de l'efficacité de leur présence auprès des personnes âgées.

qui prévoit que les crédits de la section IV du budget de la CNSA, abondant les conférences des financeurs, sont destinés à venir en soutien des aidants.

accès à ces financements dans le cadre de la conférence des financeurs. Celle-ci regroupe l'ensemble des intervenants dans ce domaine, c'est-à-dire qu'elle est au plus proche des besoins dans chaque département. Selon moi, il serait nécessaire qu'une partie de ces financements puissent être utilisés par la conférence. Je maintiens

d'un article important, qui traite des modalités d'information relatives aux proches aidants. Plusieurs de nos collègues se sont étonné que la commission des affaires sociales propose d'intégrer à la carte Vitale

mais, après avoir travaillé et y avoir réfléchi, il me semble que la carte Vitale est un vecteur de support pertinent pour ces informations. Elle rassemble certaines données pertinentes relatives au parcours de soins de la personne. Nous estimons que, à ce titre, l'identité de l'aidant y a toute sa place.

Il vise à les détecter dès que le diagnostic de la personne qu'il accompagne est posé. Cette détection permettra de leur donner une existence et de ne plus les rendre invisibles. Ainsi identifiés, ils pourront être destinataires des informations nécessaires à leur parcours d'aidant. Le duo aidant-aidé sera identifié sur les cartes Vitale des deux intéressés. Cela légitimera la place de l'aidant auprès des médecins et pharmaciens de l'aidé, par exemple. Cela évitera le « suraccident » en permettant aux services de secours de détecter que la personne qu'ils ont en charge, potentiellement incapable de s'exprimer sur le moment, apporte un soutien vital à une personne. Ainsi, l'aidé pourra être contacté et pris en charge.

alors renvoyé vers les bons services de sa commune et de son département, l'association de proximité qui pourrait l'assister dans sa vie d'aidant, et l'association la plus pertinente concernant le handicap ou la dépendance de la personne qu'elle assiste. Madame la secrétaire d'État, trop d'information tue l'information, et l'isolement tue les proches aidants ! Ils doivent être soutenus. Le guide de l'aidant, payant, de plus de cent pages, n'est pas satisfaisant, pas plus que le site internet pour les personnes âgées, qui ne propose pas de personnalisation. en proposant un parcours « clé en main » que nous pourrons accompagner efficacement les aidants. Encore une fois, je regrette l'absence de débat avec le Gouvernement qui ne propose aucun compromis.

qui préciserait, premièrement, l'organisme destinataire de la demande de la personne aidée d'intégrer le nom de son aidant au sein de sa carte Vitale, et, deuxièmement, les modalités de communication du guide du proche aidant. Quel est l'avis du Gouvernement ? Il est

L'amendement tend à élargir le champ du mécanisme, en permettant à l'aidé de figurer sur la carte Vitale de l'aidant. La mention sur la carte Vitale de l'aidant est une option intéressante. Néanmoins, cette mesure n'aura de sens que s'il peut exister un mécanisme coordonné entre les différents acteurs, notamment les professionnels médico-sociaux concernés, permettant alors de déclencher automatiquement une alerte et d'assurer une prise en charge de la personne aidée. Ce sujet est plus complexe qu'il n'y paraît. Le Gouvernement s'en

a pour objet de préciser le destinataire de la désignation de la personne de confiance d'une personne qui n'est pas admise en soins hospitaliers ou médico-sociaux. La caisse primaire d'assurance maladie n'étant pas le bon interlocuteur, il est préférable de renvoyer au médecin traitant. traitant. Quel est l'avis du Gouvernement ? L'amendement vise à modifier le destinataire de la déclaration de la personne de confiance. La caisse primaire d'assurance maladie n'étant pas le destinataire le plus pertinent, il est en effet plus judicieux que cette information soit adressée au médecin traitant ou bien, par exemple, la direction de l'établissement accueillant la personne.

des jeunes aidants, qui a un impact décisif dans le développement et l'insertion scolaire et sociale des enfants et des adolescents dans cette situation. Nous demandons un rapport au Gouvernement visant à définir les contours d'une politique publique capable d'accompagner les jeunes aidants dans leur quotidien.

Quelle égalité des chances pour ces enfants ? Près de la moitié d'entre eux affirment apporter leur aide quant à la gestion de la maison ou l'aide à la toilette, par exemple. Ces tâches quotidiennes ne sont pas sans incidence, vous le savez, sur le parcours scolaire de ces jeunes, qui se retrouvent bien souvent isolés et en décrochage. Près d'un jeune aidant sur deux est favorable à ce que l'on lui propose de l'aide pour s'occuper de la personne aidée. Trois champs d'aides sont évoqués prioritairement : des temps d'échange avec d'autres jeunes aidants, tout d'abord, l'appui d'une aide familiale, ensuite, et l'aménagement du temps scolaire ou universitaire, Ce rapport pourrait servir de base à l'intégration de mesures dédiées aux jeunes proches aidants, notamment dans le cadre de l'examen parlementaire du projet de loi pour une école de la confiance, présenté il y a peu au Conseil supérieur de l'éducation.

Mme Jocelyne Guidez, pour explication de vote. Madame la secrétaire d'État, vous ne pouvez pas mesurer mon désarroi, au moment où le Sénat s'apprête à adopter ma proposition de loi. Votre intervention, et l'expression de vos positions sur chaque amendement et chaque article montrent l'absence de réelle considération de ce gouvernement pour l'initiative parlementaire. Les aidants ne s'y tromperont pas. Vous n'avez présenté aucun amendement. Ce discours stérile n'est pas plus à la hauteur de l'enjeu que le renvoi en commission que vous aviez fait adopter au début de l'année 2018 sur le texte du député Pierre Dharréville. Malgré la présentation en juin dernier de mon initiative auprès du cabinet de Mme la ministre des solidarités et de la santé, votre collègue avouait, au début du mois d'octobre, devant mon groupe politique, qu'elle n'avait pas connaissance de son contenu. Pourtant, mes demandes de coconstruction étaient régulières. J'ai dû attendre quarante-huit heures avant la séance publique, et après que les arbitrages ont été rendus, pour que le Gouvernement me propose d'en discuter ! C'est tout bonnement de l'amateurisme et de l'irrespect pour le Parlement et, plus encore, pour les proches aidants. Ce texte sera examiné le 6 décembre prochain à l'Assemblée nationale. Oserez-vous tenir votre majorité pour qu'elle le retoque ? Oserez-vous asservir à ce point l'Assemblée nationale ? Oserez-vous expliquer à votre majorité qu'il faudra, la veille du Téléthon, refuser d'apporter le soutien, l'assistance et l'accompagnement réclamés par les proches aidants ? Oserez-vous inscrire dans le projet de loi Dépendance des mesures identiques, ayant la même finalité, que celles que vous avez balayées d'un revers de main, une année auparavant ? Oserez-vous donc, pour des raisons politiques de recherche de paternité d'un texte, ne pas entendre la détresse des proches aidants et prendre cette population en otage, au point de les laisser dans l'isolement ? Madame la secrétaire d'État, si ce projet est le vôtre, je vous souhaite bien du courage ! Du courage pour regarder en face les personnes concernées, et leurs représentants, en leur disant que vous entendez leurs préoccupations, alors que vous avez bloqué l'adoption des mesures qu'ils demandent J'en appelle donc à la raison. J'en appelle surtout à l'intime conviction des députés de votre majorité, pour qu'ils comprennent que le courage politique, c'est de se battre pour ses convictions et l'intérêt général. S'ils n'arrivent pas à nous rejoindre sur cet enjeu humain et transpartisan, alors la démocratie meurt à petit feu, car les Français, eux, soutiennent ces mesures. Ici, il ne s'agit pas d'ouvrir la boîte de Pandore, bien au contraire. Il s'agit d'apporter simplement des mesures de justice, attendues, souhaitées, désirées et salutaires. Sachez, madame la secrétaire d'État, que je suis déterminée. Trop de proches aidants attendent cette loi. Aujourd'hui, le Gouvernement n'a pas été capable de me démontrer que mes propositions n'étaient pas acceptables. Mes chers collègues, votons d'une seule voix ! La parole

l'attitude du Gouvernement, qui me rend extrêmement perplexe quant au rôle attribué à nos deux assemblées, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Le président de la commission des affaires sociales, Alain Milon, l'a dit

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, mes premiers mots seront pour féliciter ma collègue Jocelyne Guidez de sa détermination

Madame la secrétaire d'État, vous avez ici, au Sénat, la chambre de la représentation des territoires, autrement dit des élus nationaux en lien direct avec la proximité. Vous êtes témoin ce soir d'un fait exceptionnel, d'une belle unanimité : le pays entier vous parle à travers nos voix ! ( Contrairement

Leur quotidien ne ressemble pas au vôtre, celui du monde de la rationalité et de l'efficacité, où l'humanité se traite au moyen de tableurs Excel. Aussi, écoutez-les, madame la secrétaire d'État ! Écoutez ces élus qui savent, qui connaissent et qui touchent du doigt une réalité difficile à percevoir d'en haut

par votre discours introductif, madame la secrétaire d'État, j'ai souhaité dire ces quelques mots, moi, jeune sénatrice. Si l'aptitude du Sénat à créer des droits nouveaux est autorisée, alors votre discours a été particulièrement heurtant pour les élus que nous sommes. Simone de Beauvoir, que nous avons tous lue, écrivait en 1960 : « L'individu ne reçoit une dimension humaine que par la reconnaissance d'autrui ». Je crois que, aujourd'hui, la politique gouvernementale gagnerait en dimension humaine par la reconnaissance de cette

d'avoir pu prendre part longuement à ce débat, pour avoir été, comme d'autres, j'en suis certain, personnellement concerné par cette situation. Je crois que l'exemple que nous donnons aujourd'hui,

loi. C'est une lumière pour toutes les personnes en souffrance ayant besoin d'un aidant et pour les aidants eux-mêmes, qui s'investissent dans une tâche souvent très lourde.

un animateur hors pair, qui dirigeait les maisons de la culture sur mon territoire ; aujourd'hui, c'est un homme couché, qui ne reconnaît plus personne. Je me considère comme un bénévole, un proche aidant, et, lorsque je retournerai ce week-end sur mon territoire, je lui dirai que des femmes et des hommes,

Cette grande question de la scolarisation des enfants en situation de handicap est fondamentale. En effet, elle nous interroge bien au-delà du monde éducatif et du monde des accompagnants spécialisés. Elle vient questionner la capacité d'inclusion de notre société, notre rapport à ce qui est différent. En cela, la réponse des pouvoirs publics aux défis qui restent à relever sera légitimement scrutée avec attention. Je tiens, à ce titre, à remercier la présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, Catherine Morin-Desailly, d'avoir encouragé la tenue de ce débat aujourd'hui. Si le nombre d'enfants et d'adolescents en situation de handicap a beaucoup progressé au cours des dernières années, il convient toutefois de regarder par-delà les chiffres, toujours nécessaires, mais jamais suffisants.

Lorsque nous parlons d'enfants en situation de handicap, n'oublions pas qu'il existe de multiples situations en la matière : handicaps moteurs, troubles « dys », autisme, et bien d'autres encore. Très différentes, ces situations nécessitent des réponses adaptées.

et leur degré, afin qu'ils puissent accueillir le plus grand nombre d'enfants à même de bénéficier de l'enseignement ordinaire. Enfin, lorsque nous parlons de ces situations, nous nous devons aussi de prendre en compte ce qui se passe au-dehors des murs de l'école, mais en affecte la vie quotidienne. Je souhaite mentionner ici la place des familles et des aidants, tous deux essentiels à l'équilibre de l'enfant, donc à son intégration scolaire et sociale. J'ai été personnellement interpellée, dans mon département de Vendée, sur la place accordée aujourd'hui aux enfants handicapés à l'école. Ainsi, une chef d'établissement de Fontenay-le-Comte m'a alertée sur les difficultés que rencontre au quotidien le corps enseignant : manque de moyens, manque manque d'encadrement, manque d'instituts médico-éducatifs. Cette addition de manques se révèle préjudiciable à tous les enfants, avec ou sans handicap, comme aux enseignants.

Je suis sûre que nombre de mes collègues ici présents seraient facilement à même de nous présenter des exemples similaires. Cette même chef d'établissement m'a également fait part de son indignation quant à la situation salariale des AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap, vie scolaire. C'est là un point crucial de la question du handicap en milieu scolaire. En effet, comment imaginer qu'un enfant en situation de handicap puisse s'intégrer à l'école sans l'aide d'une personne spécialisée ?

les contrats à durée déterminée et les temps partiels de vingt-quatre heures hebdomadaires leur permettent difficilement d'accéder à un emploi complémentaire. Je note que le Gouvernement a engagé des mesures pour rendre plus attractif le métier d'AESH. Au demeurant, plus que d'« attraction », il devrait avant tout être question de décence. Au-delà de la question des personnels accompagnants, nous pensons qu'il convient aujourd'hui de poser les bases d'une nouvelle réflexion sur l'amélioration des structures existantes et la mise en place de solutions personnalisées. Il est en effet important d'améliorer, tant quantitativement que qualitativement, l'accompagnement des élèves handicapés. Scolariser les enfants en situation de handicap sans leur apporter le soutien dont ils ont besoin, c'est fragiliser l'ensemble du système éducatif. Il convient donc d'encourager la coopération entre les secteurs médico-social et scolaire, pour être au plus près des différents besoins de l'enfant ou de l'adolescent. Les instituts médico-éducatifs peuvent à cet égard jouer un rôle intéressant dans la mise en place de solutions personnalisées. Or la mise à disposition d'enseignants à laquelle s'est engagée l'éducation nationale se révèle très variable selon les régions et souffre d'une sous-estimation chronique des besoins. Ces structures méritent d'être mieux épaulées dans leurs missions, car elles offrent des services spécialisés et sont bien souvent une solution nécessaire à la prise en charge adaptée de l'enfant et à son épanouissement, en complément bien sûr du rôle des familles et de l'école. La stratégie du Gouvernement en matière de handicap à l'école, menée conjointement par M. Jean-Michel Blanquer et Mme Sophie Cluzel, présente certes des éléments intéressants. Ainsi, le principe de l'intégration du numérique et des dernières innovations technologiques au service de l'intégration des personnes en situation de handicap dans la société nous paraît aller dans le bon sens. De même, le coup de projecteur accordé à l'autisme permettra, je l'espère, de mieux prendre en compte les multiples facettes de cette maladie complexe et encore trop méconnue.

Vous l'aurez compris, le groupe Union Centriste sera extrêmement attentif à ce que les mesures que prendra le Gouvernement permettent une amélioration significative de la situation des élèves en situation de handicap. Nous veillerons de façon tout aussi exigeante à ce que s'améliore

poursuive le travail de contrôle qu'elle a souhaité engager au lendemain de la rentrée. Il y va, monsieur le secrétaire d'État, de la société dans laquelle nous voulons vivre. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, tous les élus ont un jour été confrontés au désarroi de parents à la recherche d'une structure d'accueil pour leur enfant porteur d'un handicap. Nous sommes évidemment très sensibles à la requête des familles, qui souhaitent le meilleur pour leurs enfants. Depuis la loi du 11 février 2005, les chiffres sont encourageants au niveau national le nombre d'enfants scolarisés en situation de handicap a plus que triplé. Le nombre d'élèves accueillis est passé d'environ 100 000 en 2006 à près de 350 000 en 2018. Dans 98 % des cas, les demandes d'accompagnement sont satisfaites. quantitativement, la réponse est bien réelle. Mais correspond-elle toujours aux attentes ? À quel sort sont livrés les 2 % qui restent sur la touche ? Nous devons analyser l'effectivité du droit à l'éducation et mesurer la portée et les limites de l'universalité des droits de l'enfant. derrière ces chiffres se cachent de grandes disparités entre les situations, mais aussi entre les départements, disparités à la mesure de la pluralité des handicaps. Les questions liées aux délais de prise en charge et à la continuité de l'accompagnement sont particulièrement saillantes. L'attente est insoutenable pour les familles, d'autant que le délai de réponse de quatre mois imposé à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est une gageure, qui dissimule de fortes disparités entre les départements. la proposition de loi examinée récemment à l'Assemblée nationale prévoyaient de diviser par deux ce délai. Sans moyen supplémentaire peut-on y parvenir ? Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un chantier prioritaire. que je connais bien. Dans mon département, la direction de l'autonomie s'est structurée pour répondre au mieux et au plus près des personnes en situation de handicap. Grâce à un partenariat et une coordination exemplaire entre les différents intervenants que sont le conseil départemental, l'éducation nationale, les collectivités et les institutions, quelque 2 400 élèves en situation de handicap ont accès à l'éducation. Certes, pour 32 enfants de notre département, seul un plan B a pu être mis en oeuvre, aucun enfant ne devant rester sans accueil. Admettons-le, certaines solutions ne sont pas à la hauteur des attentes des parents. Ce préjudice scolaire est vécu comme un préjudice moral, psychologique, voire physique. Pour toutes les situations rencontrées, l'objectif prioritaire est de favoriser l'inclusion scolaire dans le milieu dit « ordinaire ». C'est le cas de 89 % des enfants en situation de handicap en Mayenne. Pour 11 % d'entre eux, la nécessité de soins thérapeutiques n'est pas compatible avec l'inclusion scolaire. La prise en charge du handicap appelle des solutions innovantes. Dans mon département, il a été créé une unité localisée pour l'inclusion scolaire, une ULIS, intitulée « Appui en milieu ordinaire ». Les adolescents sont accueillis en CAP au sein de trois établissements scolaires différents. Un enseignant répartit son temps entre les trois établissements, afin de répondre aux difficultés rencontrées par les élèves et d'apporter les adaptations nécessaires, en lien avec les enseignants.

tel exemple illustre la nécessité de faire preuve d'imagination pour répondre à toutes les situations, dans l'intérêt exclusif de l'enfant. Les résultats intéressants obtenus en Mayenne sont le fruit d'une volonté politique de coopération efficace de tous les acteurs concernés, au bénéfice des enfants en situation de handicap. L'enfant en situation de handicap est à la fois un enfant, un patient et un élève. L'approche transversale des politiques publiques sur la question du handicap est à approfondir pour gommer les rigidités et ne pas pénaliser encore davantage les enfants et leurs familles. La recherche du bien-être de l'enfant est une quête du bonheur par la famille. Je conclurai donc par ces mots de Jacques Prévert : « Le bonheur, en partant, m'a dit qu'il reviendrait ... Que quand la colère hisserait le drapeau blanc, il comprendrait

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le droit à l'éducation pour tous les enfants est un droit fondamental. En adoptant la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la France a adopté le modèle de l'école inclusive. La scolarisation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires a ainsi connu une forte augmentation de 2006 à 2017, en passant de 100 000 enfants à plus de 320 000 enfants.

Réaliser l'École inclusive suppose le déploiement de moyens humains importants, un effort de formation de tous les personnels et l'exploitation des potentialités offertes par le numérique. Malheureusement, la réalité est tout autre. La France n'est pas un pays précurseur en la matière. Nous étions en retard, monsieur le secrétaire d'État, et nous le sommes encore. Le Conseil national d'évaluation du système scolaire fait état de fortes discriminations dans l'enseignement secondaire, dont pâtissent les élèves handicapés. Au-delà du baccalauréat, ces différences deviennent insupportables : seulement 6 % des jeunes handicapés sont diplômés de l'enseignement supérieur. Et le fossé se creuse lorsque l'étudiant vient d'un milieu défavorisé. Ce que nous observons en fin de scolarité résulte des dysfonctionnements de l'ensemble du système. L'école inclusive n'est pas encore une réalité tangible, et de nombreux défis restent à relever. Nous déplorons le manque de moyens humains et le faible niveau d'imbrication des actions en faveur de la réussite scolaire des enfants handicapés. La coopération entre éducation nationale et secteur médico-social, essentielle pour la continuité des parcours des élèves handicapés, est marginale.

situation des délais d'admission désespérément longs pour les parents d'élèves. Si les foyers les plus aisés peuvent se tourner vers des écoles privées ou scolariser leurs enfants à l'étranger, les chances pour les familles les plus précaires sont minimes. Si, au sein de l'éducation nationale, le nombre d'unités localisées et d'auxiliaires de vie scolaire pour l'inclusion scolaire augmente chaque année, leur déploiement ne s'appuie pas sur une connaissance fine des besoins, faute de statistiques et d'évaluations. Or de plus en plus d'enfants sont diagnostiqués en situation de handicap. Il s'agit notamment d'enfants présentant des troubles cognitifs spécifiques, des déficits chroniques de l'attention ou des retards de développement.

les enseignants et les accompagnants de vie scolaire ne disposent pas des compétences spécifiques nécessaires lorsqu'il s'agit de certains handicaps, tels que les troubles du spectre de l'autisme. Entre 2004 et 2014, le Conseil de l'Europe a condamné la France à cinq reprises pour violation de la Charte sociale européenne, jugeant les AVS, aujourd'hui AESH, précaires, peu formés

Le seul accès de droit à l'école de la République n'est pas suffisant. La complexité de chaque situation appelle des réponses adaptées, souples et modulables, pour sauver ces enfants de leur exil intérieur. Monsieur le secrétaire d'État, avec M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, vous avez lancé une concertation auprès du Conseil national consultatif des personnes handicapées, des parents, des organisations syndicales et des accompagnants pour rénover le dispositif d'accompagnement des élèves en situation de handicap à partir de la rentrée 2019. L'initiative est louable ; il faut espérer qu'elle débouche sur des mesures concrètes. Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, ou PIAL, sont également expérimentés dans chaque académie depuis la rentrée. Je ne doute pas qu'une évaluation sera réalisée avant la fin de l'année scolaire. Monsieur le secrétaire d'État, c'est une transformation profonde et pérenne que les parents attendent. J'entends par là des actions concrètes dignes d'un grand pays comme la France. La parole

la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapée a posé le principe d'une scolarisation en milieu ordinaire des enfants et adolescents présentant un handicap ou, à titre exceptionnel, en milieu spécialisé. Ce principe a été érigé par le Conseil d'État en obligation de résultat. Cela signifie que tout doit être mis en oeuvre pour donner un caractère « effectif » au droit à l'éducation des enfants handicapés.

une période durant laquelle ils prendront en charge un élève en situation de handicap. Je tiens également à évoquer le non-débat, à l'Assemblée nationale, de la proposition de loi d'Aurélien Pradié et la polémique qui a suivi, ce que j'ai vivement regretté. ailleurs, le Gouvernement a lancé, le 22 octobre dernier, la concertation « Ensemble pour une école inclusive », qui durera quatre mois et concernera le métier des AESH et l'accompagnement pédagogique des élèves.

Depuis 2006, le nombre d'enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a progressé sans conteste. Ainsi, de 100 000 élèves scolarisés en 2006, nous sommes passés à plus de 340 000 à la rentrée 2018. L'objectif est de parvenir à scolariser en milieu ordinaire toujours plus d'enfants en situation de handicap, mais à condition qu'ils bénéficient d'un accompagnement de qualité. En 2018, les crédits consacrés à l'accompagnement en milieu scolaire ordinaire ont considérablement augmenté.

des acteurs du handicap et de la société tout entière, pour bâtir une école réellement inclusive. Il reste du travail ! Rappelons en effet que nous manquons d'AESH, plus de 12 000 enfants n'ayant pas de solution à cette heure. De plus, il y a urgence à se pencher sur le statut des AVS et des AESH. Ce métier manque d'attractivité. Cela tient au faible nombre d'heures travaillées, à une rémunération modique, à un travail à temps partiel, à une succession de CDD et à un déficit de formation. À cet égard, je suis favorable à l'instauration d'un statut unique d'accompagnant, lequel doit devenir un véritable professionnel, formé, disposant d'un emploi stable et pérenne, rémunéré à sa juste valeur par l'éducation nationale. L'orientation prise par le Gouvernement et tendant à convertir, sur cinq ans, les contrats aidés d'AVS en contrats d'AESH, va dans le bon sens, mais n'est pas suffisante. L'accompagnement des enfants en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire ne concerne pas seulement les AESH.

Aucune structure ne doit tenir les enfants en situation de handicap éloignés de l'environnement scolaire. Toutefois, certains enfants, compte tenu de leur handicap, ne peuvent être scolarisés qu'en milieu adapté ou grâce à un accompagnement scolaire

Elle est potentiellement constitutive d'une rupture d'égalité entre enfants handicapés scolarisés et méconnaît le principe même de la compensation, qui n'a pas vocation à se substituer aux obligations incombant aux pouvoirs publics. Pour ces raisons, j'ai proposé que, quel que soit le mode de scolarisation, les accompagnants soient directement rémunérés par les pouvoirs publics. Seuls les services complémentaires comme l'aide aux devoirs pourront être financés par la PCH.

pragmatiques. Alors que les concertations sont lancées, que les groupes de travail sont mobilisés, j'espère que le Gouvernement saura s'inspirer de ses travaux, afin de faire progresser rapidement l'école inclusive. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la scolarisation des enfants en situation de handicap a fait l'objet, nous le savons, de vives polémiques ces dernières semaines à l'Assemblée nationale. Gageons que nous saurons ici, au Sénat, débattre dans le respect des uns et des autres, mais aussi- j'ose le dire -dans l'unité que ce sujet exige. Pour commencer, je voudrais saluer l'engagement quotidien de l'ensemble des acteurs- familles, associations, professionnels et enseignants -investis dans l'accueil et la prise en charge des enfants en situation de handicap dans nos établissements scolaires. Le service public d'éducation doit veiller à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Quels que soient les besoins particuliers de l'élève, c'est à l'école de s'assurer que l'environnement est adapté à sa scolarité. C'est un devoir de justice, d'équité et de solidarité. Face à ces enjeux, le débat proposé par nos collègues de l'Union Centriste, dont je salue l'initiative, intervient à un moment opportun, puisqu'il nous permet de faire un état des lieux de la rentrée 2018. Qu'en est-il ? Plus de 340 000 élèves en situation de handicap sont aujourd'hui scolarisés, c'est 20 000 élèves de plus que l'an dernier. Par ailleurs, 253 nouvelles unités localisées pour l'inclusion scolaire, les ULIS, ont été créées, dont 38 en lycée. Il faut le dire, ce progrès est le fruit d'efforts consentis depuis une dizaine d'années. Le droit à la scolarisation institué par la loi du 11 février 2005 a d'abord permis des avancées majeures, avant que le principe de l'école inclusive ne devienne en 2013 une priorité nationale. C'est ainsi que, en un peu plus de dix ans, le nombre d'élèves scolarisés en milieu ordinaire a été multiplié par La situation reste néanmoins imparfaite et inégale sur le territoire national. Aussi, j'aimerais attirer l'attention de notre Haute Assemblée sur la situation en outre-mer, où le droit à l'éducation lui-même est souvent mis à mal. En 2016, le Comité des droits de l'enfant des Nations unies y a constaté que les enfants en situation de handicap sont plus souvent scolarisés dans une classe spécialisée, en particulier en Guyane, où moins d'un élève sur six est en milieu ordinaire, et à Mayotte, où moins d'un élève sur huit Ces chiffres vont à contre-courant de la tendance observée dans l'Hexagone. En Guyane, le manque de places dans les dispositifs d'accueil de l'éducation nationale, les unités spécialisées et les structures associatives, implique que de nombreux enfants ne sont pas scolarisés Commence alors une bataille interminable pour les parents, qui n'ont souvent que leur courage pour lutter contre une nébuleuse administrative étourdissante. Pendant ce temps, l'enfant se retrouve seul, fragilisé, face au rejet que notre société lui impose. Si un effort a été consenti par le rectorat ces dernières années avec la création d'ULIS supplémentaires, la situation est particulièrement difficile pour les personnes à mobilité réduite, dont l'autonomie est fragilisée par l'inadaptation d'une grande partie de l'espace public et des transports, notamment des pirogues.

Vous verrez qu'un enfant dont le diagnostic aurait préconisé une scolarisation dans une classe spécialisée ne peut y accéder, sauf à s'éloigner dès le plus jeune âge de son foyer familial. Pourtant, vous en conviendrez, lui aussi a droit à la scolarisation. Les chiffres encourageants précédemment évoqués ne sauraient donc se suffire à eux-mêmes, tant la réussite de l'école inclusive repose également sur une amélioration qualitative des conditions d'accueil et d'accompagnement des élèves. la grande consultation, lancée ce lundi 22 octobre, va dans le bon sens. Premièrement, l'écoute attentive des familles et des associations est en effet indispensable. Ce sont elles qui vivent au quotidien le processus de scolarisation des enfants. Il est important de les soutenir, de leur donner toute leur place au sein de l'école, à travers des échanges nourris avec les équipes éducatives et l'aide de la MDPH. Deuxièmement, la transformation du métier d'accompagnant est aussi fondamentale. Pour cette rentrée, 29 000 emplois aidés et 43 000 accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH, sont mobilisés sur le terrain. pour 2019 prévoit également le financement de 12 400 nouveaux emplois d'accompagnants : 6 400 au titre de la poursuite du plan de transformation des contrats aidés et 6 000 AESH supplémentaires. Soulignons ici la volonté du Gouvernement de renforcer ces contrats, dont nous connaissons la précarité. Là encore, il nous faudra aller plus loin, en formant mieux les accompagnants, pour améliorer leurs conditions d'exercice

d'améliorer le dépistage, en particulier dans les outre-mer. Il nous faut développer les outils de diagnostic, afin d'éviter les repérages tardifs et les mauvaises orientations. Je pense à l'adaptation des outils d'évaluation au contexte plurilingue, à la visite médicale scolaire pour tous les élèves, au renforcement de la formation et à la sensibilisation des enseignants au handicap, mais aussi au développement de la PMI et du centre d'action médico-sociale précoce. Autant de pistes de travail pour adapter l'école inclusive aux réalités de nos territoires. La volonté et les initiatives sont là. Reste maintenant à faire vivre ce beau principe de l'école inclusive, grâce à une écoute attentive des familles,

si le nombre de jeunes en situation de handicap scolarisés a triplé depuis la grande loi handicap de 2005, la réalité reste insupportable pour nombre d'enfants et de familles.

jusqu'à proposer des solutions à l'étranger, notamment en Belgique. Pour d'autres familles, il ne reste plus qu'à se tourner vers l'enseignement privé, qui propose une prise en charge que le public n'offre pas toujours. Il y a surtout des enfants déscolarisés ou scolarisés à la maison, parfois pendant plusieurs années, faute de solutions adaptées, avec toutes les conséquences que cela entraîne, pour les enfants, mais aussi pour les parents- ces derniers doivent souvent cesser de travailler et vivre avec une allocation journalière de présence parentale inférieure au SMIC. Cette ambition nécessite d'accélérer la mise en accessibilité des établissements. C'est une véritable urgence, rappelée par le Conseil d'État en 2011 et par le Défenseur des droits un an plus tard. Mais les baisses successives des dotations des collectivités lorsqu'il s'agit de répondre à cet enjeu. On sait combien d'écoles, maternelles ou élémentaires, de collèges ou de lycées nécessitent encore des investissements en ce sens ! Il faut aussi évoquer les plus de 12 000 enfants qui ne relèvent pas d'une scolarisation en milieu ordinaire et qui sont en attente d'une place dans une structure adaptée, Tel est par exemple le cas du jeune Élouan, qui attend depuis 2016 une place en IME. C'est le parcours du combattant pour sa maman, qui doit multiplier les démarches pour lui en obtenir une, avant qu'il n'entre au collège, l'an prochain. si Élouan peut suivre quatre matinées à l'école élémentaire, le collège lui est formellement déconseillé. Oui, il faut créer de nouvelles places dans les établissements médico-sociaux adaptés, et il faut recruter des enseignants intervenant dans ces structures-

Vous êtes prompts à communiquer sur les 10 900 AESH supplémentaires dans les effectifs d'accompagnement à la rentrée 2018. Mais 21 000 contrats aidés ont été supprimés. Résultat, nous avons vécu, en Seine-Maritime- c'est malheureusement vrai dans beaucoup d'autres départements -, la rentrée 2018 la plus désorganisée depuis la loi de 2005.

J'évoquais la détresse des familles. Elle conduit une mère de famille d'une commune de mon territoire à menacer d'observer une grève de la faim pour espérer faire valoir les droits de son fils, Cyliann, âgé de dix ans, toujours en attente, depuis la rentrée, de l'affectation d'un AESH. tel cas n'est malheureusement pas isolé. Au problème du nombre des personnels accompagnants se conjugue la plus grande sélectivité dans l'attribution de cet accompagnement, qui en écarte certains enfants

Le choix a été fait de nier toute notion pédagogique dans l'accompagnement scolaire des élèves en situation de handicap et de réduire le niveau d'exigence lors des recrutements, au détriment des enfants accompagnés. façon, c'est presque un événement lorsque l'on daigne accorder aux accompagnants des formations leur permettant de mieux comprendre le handicap des élèves suivis, en particulier l'autisme- de nombreuses familles nous saisissent de ce problème. Des volontés diverses s'expriment pour tenter d'améliorer la situation. Et le refus même d'en débattre véritablement, constaté à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, a choqué de nombreuses familles. Nous nous réjouissons que, sur l'initiative de nos collègues du groupe Union Centriste, ce débat puisse avoir lieu aujourd'hui au Sénat.

en temps pleins tous les contrats qui peuvent l'être. En effet, les AESH ne sont pas rémunérés 1 300 euros par mois, comme cela a pu être dit : moins de 5 % d'entre elles- ce sont souvent des femmes -sont à temps complet. Nous veillerons à ce que la généralisation des accompagnements mutualisés, que les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les PIAL, vont encore favoriser, ne conduise pas à une baisse de la qualité de l'accompagnement des enfants. La solidarité nationale et l'égalité républicaine commandent que notre pays accueille et scolarise dignement les enfants et les jeunes en situation de handicap. De ce point de vue, les décisions annoncées après le comité interministériel d'aujourd'hui nous laissent sur notre faim. soit rendu possible, car ce sont en grande partie les problèmes de scolarisation, puis de qualification, qui expliquent l'importante pauvreté des personnes en situation de handicap à l'âge adulte. C'est d'ailleurs notamment en raison grande pauvreté que nous avons présenté cette semaine une proposition de loi visant à supprimer la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de l'allocation aux adultes handicapés, que trop d'entre vous, mes chers collègues, ont refusé de voter. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord me faire le porte-voix de toutes ces familles, notamment dans le Calvados, qui se mobilisent depuis la rentrée pour défendre l'accompagnement scolaire des enfants en situation de handicap.

Comment ne pas comprendre le désarroi de ces parents d'élèves handicapés qui, faute de s'être vu attribuer un AVS par l'éducation nationale, n'ont aucune solution de scolarisation, ne font bénéficier leur enfant que d'un temps d'école faible ou doivent patienter sur les listes d'attente des établissements spécialisés ? En 2018, en France, le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, devrait être un droit effectif. C'est une question de justice sociale et de solidarité. Le Gouvernement a lancé, lundi dernier, une concertation visant à « rénover les dispositifs d'accompagnement pour les écoliers ayant des besoins spécifiques tout au long de leur scolarité ». Des sujets centraux comme ceux de la formation des enseignants ou du statut des accompagnants d'élèves handicapés vont être abordés. C'est une bonne chose, et je salue cette volonté. En même temps, je regrette qu'il n'ait pas été possible de débattre, très récemment encore à l'Assemblée nationale- cela a été évoqué -, d'une proposition de loi relative à l'inclusion des élèves en situation de handicap. Ce soir, je souhaite profiter de ce débat pour vous alerter, monsieur le secrétaire d'État, sur la nécessaire remise à plat des dispositifs d'accompagnement existants, au regard de la situation actuelle des enfants atteints de troubles spécifiques du langage et des apprentissages,

de l'adoption de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013 et de la publication de la circulaire du 22 janvier 2015, un plan d'accompagnement personnalisé, ou PAP, peut être proposé aux enfants présentant des troubles des apprentissages. Dans les faits, ce dispositif se substitue à celui du projet personnalisé de scolarisation, ou PPS. Les enfants « dys » et TDAH sont donc placés en dehors du champ de la politique du handicap et privés ainsi du bénéfice de l'accès à un certain nombre d'aides et de droits.

Surtout, il est basé sur la notion peu claire et approximative de « difficultés scolaires » et n'est donc pas adapté à des enfants en situation de handicap, « dys ces troubles nécessitant une connaissance fine du tableau cognitif de l'enfant, qui permettra d'identifier les fonctions déficitaires mais aussi et surtout celles qui sont préservées. des personnes handicapées, renvoient les « dys » et TDAH vers le PAP, y compris lorsque les troubles sont importants et multiples et lorsque les dossiers de demande d'aide des familles sont complets et fondés. Ainsi écartés du champ du handicap et des mesures dédiées, les familles ne peuvent se voir attribuer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, allocation compensatoire qui permet de financer les indispensables bilans complémentaires et d'aider à faire face aux coûts des rééducations non remboursables par la sécurité sociale.

Monsieur le secrétaire d'État, pour toutes ces raisons, il est urgent d'entendre les arguments de ces familles ainsi que des professionnels, qu'ils soient orthophonistes, psychomotriciens ou ergothérapeutes.

Je souhaite donc que la concertation que vous avez lancée lundi dernier mette définitivement un terme à cette situation hautement préjudiciable aux enfants atteints de troubles spécifiques du langage et des apprentissages, « dys », TDAH et à leurs familles. La parole

le 11 octobre dernier à l'Assemblée nationale. Vous le savez, notre groupe, le RDSE, est particulièrement attaché à la qualité du débat parlementaire ; j'espère que le Sénat, dans sa grande sagesse, mènera la discussion à son terme et la fera prospérer sous forme législative. En avril dernier, le Gouvernement a annoncé vouloir mettre l'accent sur le diagnostic et sur la scolarisation des enfants dans le cadre du quatrième plan Autisme, qui a pour objectif le triplement du nombre d'unités d'enseignement en maternelle, la création de cent postes d'enseignants spécialisés,

Il reste donc à trouver une stratégie plus globale associant les différents acteurs du soin et de la scolarisation pour faire face à la demande croissante des élèves en situation de handicap, qui reste, à ce jour, non entièrement satisfaite. Toutefois, je profite de cette tribune pour féliciter le service d'éducation spéciale et de soins à domicile pour le travail accompli à Saint-Martin

Néanmoins, un travail important doit être conduit pour dépister plus efficacement et surtout plus précocement un certain nombre de troubles, tels l'autisme ou la dyslexie ; cela passe nécessairement par une meilleure sensibilisation des professionnels de santé, des parents et de la société. il n'y a pas qu'à Saint-Martin que ce travail doit se poursuivre : malgré le développement continu de l'aide mutualisée et de la création d'ULIS, entre 30 et 1 500 élèves par département attendent toujours un accompagnement. Aujourd'hui, malgré plusieurs plans Autisme et plans quinquennaux concernant le handicap, les contraintes budgétaires ne nous permettent pas de rattraper le retard accumulé. Un rapport sénatorial de décembre 2016 nous enseignait par exemple que, en 2015, quelque 1 500 enfants en situation de handicap étaient pris en charge en Belgique et conventionnés par l'assurance maladie. Faut-il voir dans cette sous-traitance le signe de défaillances en matière de planification ?

en établissements spécialisés soient scolarisés à l'école. Mais ce volontarisme nécessitera une étroite articulation entre tous les services. De ce point de vue, je porte à votre attention trois interrogations. quelle est votre stratégie pour opérer ce grand changement, associant les différents acteurs du soin et de la scolarisation et décloisonnant les interventions et les dispositifs, pour faire de l'école ce lieu institutionnel effectivement central de la prise en compte des besoins de tous les enfants ?

Les unités d'enseignement externalisées et les unités de soins mobiles devraient pouvoir être décuplées et pilotées au sein d'une plateforme de services à l'échelon départemental. L'urgence est aussi de répondre à la situation de ceux que nous appelons les « invisibles de l'éducation nationale », à savoir les auxiliaires de vie scolaire, les AVS, et les accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH.

ailleurs, comment lutter contre la forte inégalité des situations entre les territoires, les solutions et les services proposés aux enfants en situation de handicap variant selon les établissements ? Enfin, le Gouvernement a annoncé l'ouverture de 250 ULIS à l'horizon 2022. Mais, dans un récent rapport, l'IGAS a précisé que, au rythme actuel de progression du nombre d'enfants devant être pris en charge en ULIS, il faudrait ouvrir non pas 50 unités supplémentaires par an d'ici 2022, mais 240 en moyenne. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la loi de 2005 a marqué un tournant décisif en direction de l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap- c'est indéniable. Les effets qu'elle a produits apparaissent extrêmement positifs. Cependant, de nombreux défis subsistent sur le chemin qui doit permettre à l'école d'instruire et d'éduquer tous les enfants et adolescents en situation de handicap, sans distinction aucune.

Une fois accepté par la famille, ce PPS s'impose aux établissements scolaires, donc aux enseignants, lesquels, en milieu ordinaire, n'ont pas été impliqués dans le projet.

là où l'éducation nationale est fortement présente et impliquée dans les équipes des CDAPH. En revanche, les enseignants, eux, restent démunis

Convenons que le sujet n'est pas simple et que la feuille de route du Gouvernement, qui va dans le bon sens, rencontre une adhésion certaine de la part des acteurs impliqués. Pour ma part, je soutiens la création de postes d'AESH

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, de toutes les révolutions qu'a connues notre pays depuis 1789, la plus heureuse et peut-être la plus importante est la « révolution scolaire C'est avec les lois dites « Jules Ferry » instaurant la gratuité, la laïcité, mais aussi l'obligation de la scolarité, dans les années 1880, que s'est réellement développé et démocratisé l'enseignement, d'abord au niveau primaire. La République offrait ainsi à tous ses enfants l'accès au savoir, leur permettant d'espérer une progression sociale à travers la réussite scolaire et la reconnaissance des mérites de chacun. À tous ses enfants, dis-je - Au fil des décennies et des Républiques, l'esprit desdites lois a été décliné et complété, avec une démocratisation de l'accès au collège, puis au lycée, enfin à l'université. Mais cette belle oeuvre de diffusion du savoir dans toutes les couches de la société a longtemps, trop longtemps, oublié les enfants en situation de handicap.

beaucoup pour accueillir ces élèves différents et pour les intégrer au mieux au sein des classes. L'instauration, en 2000, des auxiliaires de vie scolaire, AVS, désormais accompagnants des élèves en situation de handicap, AESH, a été une étape charnière. Aujourd'hui, il est d'ailleurs difficilement envisageable d'imaginer la scolarisation des enfants handicapés sans l'aide des AESH., bien des parents, mais aussi des enseignants, déplorent le nombre insuffisant nombre insuffisant de ces personnels dont le statut et la formation sont à préciser. La récente rentrée scolaire a d'ailleurs eu son lot de déceptions et de mécontentements, avec de nombreux enfants sans AESH, mais aussi

Afin d'améliorer encore cette insertion des élèves en situation de handicap au coeur des classes « traditionnelles », il pourrait être précieux de permettre aux enseignants de mieux appréhender et comprendre les difficultés spécifiques et toujours particulières de ces enfants. En effet, le code de l'éducation prévoit très précisément, dans son article L. 721-2, que « les écoles supérieures du professorat et de l'éducation [ ...] organisent des formations de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations,

Aussi pourrait-il être pertinent et formateur d'inclure dans le cursus des futurs professeurs une période consacrée exclusivement à l'accompagnement d'élèves handicapés. C'est d'ailleurs l'objet d'une proposition de loi que j'ai déposée le 13 juin dernier, qu'a évoquée mon collègue et ami Philippe Mouiller et qui a été cosignée par près de cent sénateurs siégeant sur tous les travées, ou presque, de l'hémicycle. L'idée est simple : durant sa formation, l'apprenti enseignant remplirait pour plusieurs semaines- pourquoi pas pour un mois, voire pour un trimestre ? -la même mission qu'un AESH, afin de bien intégrer les attentes et les besoins de l'élève qui se trouve sous sa responsabilité. L'expérience ainsi acquise serait évidemment utile aux futurs « maîtres » lorsqu'ils auront à gérer des effectifs comprenant un ou plusieurs élèves en situation de handicap, que ces derniers soient ou non « tutorés » par un AESH. L'autre intérêt de ce dispositif serait de permettre la prise en charge individuelle d'enfants handicapés en bien plus grand nombre qu'aujourd'hui. Le coût d'une telle mesure serait par ailleurs très raisonnable. D'autres pistes sont aussi à creuser dans le cadre de la formation continue des enseignants titulaires. C'est une question d'imagination, mais surtout de volonté gouvernementale. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, s'il est essentiel de renforcer les effectifs d'AESH, ainsi que d'améliorer leur statut et leur formation en les professionnalisant, il est tout aussi indispensable de former les enseignants eux-mêmes à cet accueil des élèves en situation de handicap. C'est au soin qu'elle apporte aux plus fragiles qu'on mesure la grandeur et la dignité d'une société. En matière de scolarisation des élèves en situation de handicap, des progrès ont été réalisés,

Jasmin. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens à remercier mes collègues d'avoir inscrit ce sujet à l'ordre du jour de nos travaux, tant cette problématique est importante à nos yeux.

de nombreux enfants et adolescents qu'on ne peut se résoudre à laisser hors de l'institution scolaire. L'inclusion sociale des enfants atteints de handicap constitue donc une absolue nécessité. nécessité. En 2002 déjà, interpellai-je la communauté éducative, au sein du conseil de l'éducation nationale de la préfecture de Guadeloupe, sur les problématiques liées au handicap. En 2004, en ma qualité de présidente d'une fédération de parents d'élèves, je fus à l'initiative de la mise en place d'une classe dédiée

Aujourd'hui, monsieur le secrétaire d'État, un inventaire statistique et un état des lieux précis portant sur les différents dispositifs existants serait salutaire, afin d'adapter au mieux le projet de loi annoncé par votre gouvernement à la réalité des besoins des enfants, des parents, des associations et des territoires.

Face à l'augmentation des besoins, il devient indispensable de repenser la scolarité de ces enfants comme un parcours continu d'apprentissage personnalisé, à la fois sur le temps scolaire et sur le temps péri-périscolaire. Cette transformation passe par une mobilisation de tous : l'État bien sûr, les collectivités locales, les conférences régionales de santé et de l'autonomie, les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les maisons départementales du handicap, ainsi que tous les acteurs médico-sociaux libéraux et associatifs, avec le soutien des familles, afin de favoriser une prise en charge effectivement transversale et inclusive. Je préconise des personnels de l'éducation, les enseignants et les non enseignants, tels que les ATSEM, les animateurs, les personnels d'orientation, plus nombreux et et mieux formés, grâce à des modules obligatoires sur le handicap dans le cadre de leur formation initiale et continue, comme l'apprentissage des fondamentaux de la langue des signes, par exemple. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap doivent disposer d'un statut unifié et être mieux rémunérés, avec un référentiel des métiers clair et mieux valorisé. un accompagnement des collectivités locales sur l'accessibilité du bâti et des outils pédagogiques, par exemple, pour les élèves du second degré, des espaces de lecture

de recevoir les messages d'alerte et d'urgence. Il faut mettre en place un référentiel national applicable sur l'ensemble du territoire de la République, notamment pour les aménagements nécessaires pour le passage des diplômes et examens par des personnes en situation de handicap. Pour favoriser l'utilisation de l'alternance et de l'apprentissage dans les différentes branches professionnelles, pour les jeunes en situation de handicap, il serait également utile de renforcer l'accompagnement spécifique pour les entreprises

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le 22 mai dernier, en prévision de la rentrée scolaire 2017-2018, j'ai interrogé le Gouvernement sur la situation précaire des AVS et des AESH.

Faudra-t-il qu'un drame survienne pour que, enfin, l'on considère ces personnels ? « Ensemble pour une école de la confiance », déclarez-vous ... Oui, nous sommes tous tout à fait d'accord

Dois-je rappeler que le nombre des enfants en situation de handicap est en constante augmentation ? Le recrutement sera encouragé, comme le prévoit le décret de juillet 2018. Sera-t-il suffisant pour contenter toutes les demandes des parents ? Le salaire des personnels sera-t-il revalorisé ? Je le souligne, le salaire moyen d'un assistant est de 700 euros par mois. Ces personnels sont mal rémunérés, en sous-effectifs et en manque de reconnaissance, sans parler de l'absence de formation préalable pour la plupart d'entre eux. Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite vous soumettre un cas concret rencontré en Aquitaine, mais il en existe évidemment bien d'autres ailleurs. À la fin du mois de septembre dernier, un nombre important de personnels en renouvellement de CDD ou bénéficiant d'un contrat nouveau n'ont pas touché l'intégralité de leur salaire. Le rectorat de Bordeaux invoque une transmission tardive de leur dossier, ce qui est faux ! Les salaires ne sont pas versés intégralement par l'éducation nationale. Certains accompagnants, sans être avertis, n'ont perçu à la mi-octobre que 70 % de leur salaire de septembre, le reste devant être versé avec le salaire d'octobre. Ils n'ont toujours rien reçu à ce jour. sera-t-il ? Au-delà de la situation financière difficile que vivent la majorité des AVS ou AESH, se pose le problème de leur statut. Les contrats existants ne pérennisent pas les emplois et fragilisent la relation de confiance qui s'établit entre les enfants, les enseignants et la famille. Les enseignants reconnaissent eux-mêmes que, sans ces accompagnants, il leur serait difficile de gérer une classe accueillant un enfant handicapé.

sans doute en raison du mécontentement exprimé à la rentrée par les parents des élèves concernés, le Gouvernement esquisse un plan en faveur des AVS et des AESH sur la base de l'expérimentation de pôles inclusifs d'accompagnement localisés, à coup d'annonces dans la presse.

de leur offrir le meilleur environnement scolaire possible ? Si nous devons, nous tous ici réunis, respecter un des principes fondateurs de la République, l'école pour tous, il serait stupéfiant que vous ne le respectiez pas aussi.

peu biaisée. À la rentrée 2018, quelque 29 000 emplois aidés et 43 041 AESH en équivalents temps plein accompagnaient les élèves en situation de handicap. Je veux le rappeler, aucun contrat aidé dédié à l'accompagnement du handicap

Ces chiffres traduisent concrètement la volonté du Gouvernement d'offrir un statut stable et pérenne aux accompagnants. La pérennité passe également par l'amélioration de la formation des professeurs et des accompagnants.

tous les enseignants bénéficient dans le cadre de leur formation de modules sur l'accueil des élèves en situation de handicap. Cet engagement, qui est très fort, sera au coeur de la réforme. La hausse de la scolarisation des élèves en situation de handicap est une réussite collective. Elle implique désormais une évolution de la fonction d'accompagnant de ces élèves.